Monsieur le président,

La séance est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du jeudi 24 janvier 2019 a été publié sur le site internet du Sénat.

L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (projet n° 28, texte de la commission spéciale

je suis particulièrement heureux de vous présenter en séance ce projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, et je me réjouis par avance, avec ma secrétaire d'État Agnès Pannier-Runacher, des débats constructifs que nous allons avoir dans les jours à venir. Ce projet de loi PACTE, c'est dix-huit mois de dialogue pour offrir de véritables solutions, permettant à nos entreprises de grandir, d'investir, d'innover, d'embaucher

des échanges que nous avons eus avec les entrepreneurs, les salariés, les fédérations professionnelles, les organisations syndicales. Dialogue avec les parlementaires, bien sûr.

Je voudrais tout particulièrement remercier la présidente de la commission spéciale, Catherine Fournier, le rapporteur sur le chapitre I, Élisabeth Lamure, le rapporteur sur le chapitre II, Jean-François Husson, et le rapporteur sur les chapitres III et IV, Michel Canevet, pour le travail remarquable qu'ils ont réalisé afin d'étudier les possibilités d'amélioration du texte.

Ces blocages, nous allons, tous ensemble, les lever ! Cela passe par la simplification. Nous nous sommes fait une spécialité, en France, de la complexité administrative, et celle-ci est

Parmi ces simplifications, il est une mesure emblématique, celle qui, à mon sens, est la plus à même de permettre à nos PME de grandir

La modification des seuils est décisive pour libérer la création de dizaines de milliers d'emplois dans notre pays. Je suis donc prêt à étudier, de manière ouverte et constructive, les propositions d'amélioration que vous ferez sur ce thème. L'innovation, ensuite : c'est la condition de la compétitivité de nos entreprises. Sur ce sujet, soyons lucides. Nos entreprises ont pris du retard en matière de digitalisation

Tous les moyens de financement que nous allons mettre en place pour faciliter les expérimentations, donner plus de transparence aux, les ICO, construire des ponts entre la recherche publique et l'entreprise vont nous permettre de développer l'innovation et de lever, là aussi, certains freins incompréhensibles du lien entre innovation et entrepreneuriat. Ainsi, comment accepter que l'on ait bridé, à ce point, la possibilité, pour un chercheur, de travailler dans une entreprise ? Pourquoi a-t-on empêché un chercheur de posséder des participations dans une entreprise et de les conserver après son retour dans le monde de la recherche ? Levons ces freins et ces obstacles, qui ont empêché le le talent français de s'exprimer au niveau qui est le sien ! La justice, enfin, car le travail doit payer. Le travail doit payer en France

sont la première condition de la réussite d'une entreprise. Il est légitime que, lorsqu'une entreprise réussit, ses salariés en soient récompensés, l'intéressement ou la participation.

faut aussi remédier à la faiblesse actuelle du statut de conjoint collaborateur pour les indépendants, qu'ils soient artisans, commerçants ou professions libérales. Un quart des indépendants travaillent avec leur conjoint, dans le cadre d'un temps partiel ou d'un temps complet. Or près d'un tiers de ces conjoints,

ces grandes lignes font consensus et je salue le dialogue constructif que nous avons engagé avec les rapporteurs sur les différents volets de ce projet de loi. Il va dans l'intérêt de l'économie française, l'intérêt des PME que ce texte entre en vigueur le plus vite possible. Il est attendu par les chefs d'entreprise, par les PME, par les commerçants, qui savent que ce texte libérera les capacités d'embauche, d'investissement et d'innovation. Je vous propose donc que nous essayions de l'adopter dans les plus brefs délais, en trouvant un accord entre nous sur ces grandes lignes. Nous avons d'ailleurs, grâce au travail des rapporteurs, beaucoup progressé sur un certain nombre de sujets. Je pense à la redéfinition de l'objet social de l'entreprise dans le code civil, à la réforme des seuils d'audit pour les commissaires aux comptes, à la réforme de l'épargne retraite, retraite, à la fusion entre La Poste et CNP Assurances, qui donne naissance à un grand ensemble financier public, au service des territoires auxquels vous êtes profondément attachés. Vous avez formulé des propositions pour améliorer le texte, notamment celle qui vise à renforcer la présence des élus des territoires au conseil d'administration de La Poste. Je suis favorable à tout ce qui permettra d'obtenir un texte sorti du Sénat meilleur qu'il n'y était entré. J'en viens à un certain nombre de sujets sur lesquels vous avez marqué votre sensibilité. Premier sujet d'attention particulière, les territoires. qualité d'élus de nos territoires, vous m'avez signalé l'importance que vous attachez à la présence des acteurs économiques dans les territoires, notamment les chambres de

à les renforcer, en proposant un nouveau modèle de financement, plus solide que celui de la taxe affectée. Il y a là un enjeu de transformation. Tous les présidents de CCI et de CMA que j'ai rencontrés sont parfaitement lucides sur ce sujet. Il faut de nouvelles modalités de financement, de nouvelles modalités de recrutement et de nouvelles modalités d'organisation des chambres consulaires : c'est ce qui vous est proposé. J'attacherai une importance toute particulière aux chambres de commerce des territoires les plus ruraux, là où, peut-être, elles sont les plus utiles,

d'opposition entre nous- mais cela fait partie du débat démocratique -, les cessions d'actifs dans Aéroports de Paris, la Française des jeux et Engie. Vous me permettrez de prendre un peu de temps pour expliquer les choix politiques et économiques qui sous-tendent la proposition que nous vous faisons. Je ferai un premier constat, à mes yeux le plus important : ce sont les innovations de rupture qui tirent désormais l'économie mondiale. Ces innovations de rupture feront la différence entre les économies qui réussiront et celles qui échoueront.

feront la différence entre les nations qui resteront debout et celles qui seront soumises, entre les nations qui demeureront souveraines et productrices et celles qui n'auront plus d'autre choix que de devenir vassales et clientes de la Chine et des États-Unis.

Tous ceux qui nous parlent d'industrie matin, midi et soir- à juste titre, parce que nous voulons reconquérir notre place industrielle dans le monde -ne doivent jamais oublier qu'elle coûte cher. Ce sont des équipements lourds et des investissements stratégiques. Oui, il faut de l'argent pour gagner la bataille de l'innovation. Nous avons besoin de conditions financières compétitives. Pour cela, il nous faut des fonds propres, car l'argent de la dette

Le prélèvement forfaitaire unique et l'allégement de la fiscalité sur le capital doivent nous permettre de financer nos entreprises et de ! ... que nous avons faits sur le crédit d'impôt recherche, le CIR, la décision que nous avons prise de donner aux entreprises deux années de suramortissement pour qu'elles puissent acheter des robots et se digitaliser sont la condition du redressement de notre pays.

échéance, au taux de 25 %. Il n'a jamais été question, et il ne le sera jamais, de remettre en cause cette trajectoire de l'impôt sur les sociétés, qui est une condition clé de l'attractivité du territoire français et du développement de nos entreprises. La troisième arme pour gagner cette bataille de l'innovation, après celle des compétences, après celle du financement, c'est la protection. Nous n'investissons pas dans les nouvelles technologies pour nous faire piller par nos partenaires ou par nos voisins. Là, je suis d'accord ! Il faut donc mieux nous protéger, comme le font, d'ailleurs, les États-Unis, la Chine et toutes les grandes puissances de la planète.

Le règlement européen sur le des investissements étrangers en Europe sera aussi une étape majeure. Il marque une véritable prise de conscience par l'Europe de la nécessité de protéger ses technologies.

comme l'autonomie des véhicules. Nous ne pouvons et nous ne voulons prendre aucun risque en la matière. Il ne s'agit en aucun cas de cibler un équipementier en particulier, mais nous nous doterons des moyens de protéger les données sensibles dans le cadre du déploiement de la 5G

Elles nous permettront de financer des technologies qui garantiront, demain, notre souveraineté. L'un des premiers défis que nous allons relever au travers de ce fonds pour l'innovation de rupture, c'est la recherche sur les batteries électriques. me rendrai dans quelques jours à Berlin pour rencontrer mon homologue allemand, Peter Altmaier. Nous allons mettre en place, à la suite de l'accord entre le Président de la République et la Chancelière, une filière de

Sans le financement du fonds pour l'innovation de rupture, on ne peut envisager la mise en place de cette filière de batteries, qui garantit notre autonomie, notre souveraineté, notre liberté et notre puissance économique. j'entends bien sûr les inquiétudes, les critiques qui se sont exprimées dans les rangs de votre assemblée. J'entends les comparaisons, un peu rapides, qui sont faites avec le précédent des autoroutes. Je veux vous dire que nous avons tiré toutes les conséquences de ces précédents. Des erreurs ont été faites, nous ne referons pas les mêmes. Nous garantirons les intérêts à long terme de nos compatriotes et de l'État ; nous renforcerons le cadre de régulation pour éviter que les futurs acteurs présents au capital n'abusent de leur position.

Le cadre de régulation sera plus strict après cette opération qu'il ne l'était avant. Premier point

des infrastructures d'Aéroports de Paris, des pistes et du foncier, c'est que 49 % de propriétaires privés ont un accès illimité, à vie et au-delà,

Une ligne dans la loi aurait suffi à faire cette privatisation ! Jamais, je dis bien jamais, je n'ai envisagé cette solution de facilité qui ne préserverait pas les intérêts de l'État, nos intérêts patrimoniaux et les intérêts de nos compatriotes. Ne parlons pas de privatisation sèche là où il n'en a jamais été question et là où nous ne l'avons jamais envisagé ! Grâce à cette opération, ! ... va pouvoir retrouver au bout de soixante-dix ans la pleine propriété de ces actifs, qui appartiennent aujourd'hui, je le rappelle, pour une durée illimitée, à hauteur de 49 % à des acteurs privés.

ou trop aléatoire, alors qu'il n'est pas en mesure de le faire aujourd'hui. C'est bien pour cela que je vous dis que le cahier des charges permet de renforcer le contrôle de l'État par rapport à la situation précédente. L'Assemblée nationale a renforcé ce cahier des charges, notamment des propositions du groupe socialiste visant à inclure dans celui-ci le statut des personnels et la question de l'emploi.

? Je compte sur le sens des responsabilités et sur la sagesse des sénateurs pour savoir reconnaître que les frontières resteront les frontières, que le contrôle restera aux mains de l'État, que les douanes resteront les douanes et qu'on comptera toujours autant de policiers aux frontières pour contrôler l'arrivée des personnes et des biens ! Avant ou après l'opération, rien ne change à l'exercice des missions souveraines de l'État. Rien, absolument rien ! Ne jouons pas avec les peurs des Français ! Donc, ne le faites pas ! Je connais suffisamment la sagesse de cette assemblée pour savoir qu'elle reconnaîtra que les enjeux de souveraineté ne sont en aucun cas modifiés par cette opération. Alors, j'entends aussi ceux qui me disent : « Il vaudrait peut-être mieux continuer à toucher des dividendes que de placer l'argent dans un fonds : cela nous rapporterait exactement la même chose. » Mais c'est faux ! Ah bon ? Il se trouve que, à ce jour, les dividendes sont élevés. Mais, en 2008, ils n'existaient pas ! Si vous voulez financer l'innovation de rupture par de l'argent qui est disponible une année, mais qui ne l'est pas l'année suivante, je vous souhaite bien du courage ! C'est comme cela qu'on empêche notre pays de gagner la bataille de l'innovation, de l'investissement et des nouvelles technologies. Alors on me dit : « ADP, c'est une infrastructure absolument stratégique. » Ce qui est stratégique, ce sont les redevances-

des hôtels et des boutiques de luxe. Si vous estimez que le rôle de l'État est de gérer des hôtels et des boutiques de luxe, telle n'est pas ma conception. Je considère Je considère au contraire que cette opération est un moyen de développer Aéroports de Paris, que c'est un moyen d'en faire le leader mondial en matière aéroportuaire, que c'est un moyen d'investir massivement dans les technologies critiques, qui feront la souveraineté et la liberté de la France. Je considère que cette opération doit nous permettre de trancher une bonne fois pour toutes un débat qui est essentiel pour la France : qu'est-ce que font les entreprises et qu'est-ce que fait l'État ? qu'est-ce que fait le service public et qu'est-ce que fait le secteur privé ? Je considère que c'est le rôle du secteur privé de gérer des affaires commerciales, comme il le fera pour ADP, et je considère que le rôle de l'État est de se recentrer sur ses missions stratégiques de souveraineté, de protection des Français, de santé et d'éducation. C'est aussi le choix qui vous est proposé au travers de ces cessions d'actifs. voilà les quelques éléments que je voulais vous présenter, en prenant le temps nécessaire pour vous expliquer le sens de ces cessions d'actifs et le sens de ce projet de loi PACTE. Vous le voyez bien, l'enjeu dépasse ce simple texte : l'enjeu, c'est de savoir

libres, dont les carcans liés aux seuils, à la complexité administrative, aux enregistrements seront enfin supprimés. Nous voulons une économie qui rémunère bien les salariés : c'est l'intéressement, c'est la participation. Illusionniste ! Ce sont les choix qui ont été faits par cette majorité depuis plusieurs mois. Nous voulons une économie dans laquelle les rôles respectifs de l'État et de l'entreprise sont enfin clarifiés. Nous ne voulons plus d'un État qui se mêle de tout, de ce qui ne le concerne pas nécessairement, pour laisser aux entreprises la capacité de développer les talents considérables de notre nation et de nos entrepreneurs. Nous voulons une économie qui innove, une économie qui retrouve le génie français, qui est un génie de créativité, de technologie, de recherche, de puissance intellectuelle, qui a toujours fait dans notre histoire notre force. Ce qu'il y a derrière PACTE, c'est tout simplement la capacité à donner de la prospérité à tous les Français et à tous les territoires. Je me réjouis d'avoir ce débat sur l'avenir de notre économie avec vous ! La parole

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi que très attendu par les entreprises et l'Assemblée nationale y a ajouté des mesures intéressantes. Les trois rapporteurs que nous sommes ont donc abordé ce texte dans un esprit constructif.

De 73 articles au départ, le texte est passé à 196 articles à la suite de son examen par l'Assemblée nationale, c'est-à-dire 123 articles sans étude d'impact. Dans un esprit de modération, notre commission a supprimé 37 articles et adopté un texte de 174 articles au final. telle ampleur peut donner l'impression d'un champ trop vaste, avec des sujets parfois insuffisamment approfondis. On peut ainsi déplorer un manque de préparation sur certains dispositifs, qui conduit le Gouvernement à nous présenter aujourd'hui de nouveaux amendements, à l'exemple du registre unique des entreprises. Dans cette diversité de sujets, certaines mesures sont parfois bien modestes au regard des ambitions affichées : je pense, par exemple, à celles qui concernent le rebond des entrepreneurs. L'envie d'aller plus loin n'a donc pas manqué, toujours au service de nos entreprises.

compte tenu de la concentration des nouvelles obligations sur le seuil de 50 salariés résultant du projet de loi et de l'inadéquation de ce seuil avec la croissance des entreprises. La commission spéciale a approuvé les nouvelles règles d'appréciation et de franchissement des seuils s'appliquant en matière fiscale et sociale. La commission spéciale a accepté, non sans regret, l'économie générale de la réforme du contrôle légal des comptes, consistant à relever les seuils de contrôle obligatoire par un commissaire aux comptes au niveau prévu par le droit européen. Il n'est pas certain que cette réforme soit sans effet négatif sur la sécurité financière de nos entreprises, sans même parler de l'impact très lourd sur la profession et sur son implantation dans nos territoires, au profit de grands cabinets le plus souvent anglo-saxons. La commission spéciale a repoussé l'entrée en vigueur de cette réforme à 2021, pour permettre à la profession de se réorganiser et de développer de nouveaux services aux entreprises, en dehors du contrôle obligatoire, en particulier le nouvel audit simplifié pour les petites entreprises prévu par le projet de loi. Elle a également veillé à ce qu'un contrôle suffisant soit exercé dans les groupes. Concernant la mutation du réseau des chambres de commerce et d'industrie, la commission spéciale a voulu sécuriser la situation des personnels, y compris en matière d'assurance chômage, et faciliter les restructurations des établissements et des entités du réseau, notamment avec la suppression des guichets des centres de formalités des entreprises dès 2021 et le maintien d'une politique de péréquation budgétaire entre les chambres. défendant les actions de proximité en faveur des artisans, la commission spéciale a refusé la régionalisation forcée du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat telle qu'elle était proposée dans le texte adopté par l'Assemblée nationale, se réservant toutefois la possibilité d'y revenir- nous verrons cela sans doute dès demain matin. Pour autant, elle a encouragé la mutualisation des actions des réseaux consulaires, en préservant leur pleine liberté dans ce domaine. S'agissant des brevets, la commission spéciale a approuvé les mesures prévues par le texte, de nature à améliorer la compétitivité des entreprises, spécialement les PME, en protégeant leur capacité d'innovation. En particulier, le brevet français est renforcé afin d'en faire un vrai outil de lutte contre la contrefaçon et de valorisation du capital immatériel. L'instauration d'une procédure administrative d'opposition aux brevets sera très utile pour les entreprises, en leur permettant de mieux défendre leurs titres de propriété sans avoir à emprunter la voie judiciaire, plus longue et plus coûteuse. Enfin, la commission spéciale a approuvé le renforcement du dispositif de contrôle des investissements étrangers prévu par le texte. Alors que les entreprises françaises sont particulièrement attractives et bénéficient d'un niveau élevé d'investissement en provenance de pays tiers, il est nécessaire de protéger nos activités stratégiques. Les mesures prévues ajoutent de nouveaux outils de contrôle et de dialogue, prévoient une information régulière du Parlement et du public et renforcent les sanctions.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le défi est de taille : 200 secondes pour parler de 196 articles ! Merci au Sénat d'avoir allégé de 37

La commission spéciale, sous l'autorité bienveillante de sa présidente, a d'ailleurs conforté les dispositions visant à améliorer et à diversifier les financements des entreprises, tout en adoptant de nombreux aménagements. Trois objectifs nous ont guidés : compléter les réformes, lorsque nous avons estimé que le projet de loi « s'arrêtait au milieu du gué »- je pense par exemple à la réforme du PEA-PME garantir leur effectivité, face à des dispositions trop souvent mal ajustées et/ou adoptées dans la précipitation examiner ces réformes à travers d'autres prismes que le seul financement de l'économie. À titre d'exemple, si les levées de fonds en crypto-actifs constituent une nouvelle forme de financement pour les start-up et un facteur d'attractivité pour la place de Paris, la commission spéciale a significativement renforcé le cadre de régulation proposé afin de protéger les épargnants, notamment individuels, des « arnaques » et de veiller à ce que ces nouveaux outils ne constituent pas un vecteur de blanchiment ou de financement du terrorisme. S'agissant de l'épargne retraite, la commission spéciale s'est attachée à mieux prendre en compte les enjeux liés à la dépendance, tout en encourageant fiscalement la sortie en rente, plus protectrice pour nos aînés.

Cela m'amène à évoquer brièvement les mesures visant à faire évoluer le capital des entreprises publiques, au premier rang desquelles figurent la privatisation de la Française des jeux et celle d'Aéroports de Paris. S'agissant de la Française des jeux, la commission spéciale a considéré que le Gouvernement demandait aux parlementaires de lui signer un véritable « chèque en blanc », en l'absence de définition des modalités de la future régulation et, notamment, de la fiscalité. Compte tenu des enjeux majeurs pour les finances publiques, mais aussi pour la santé publique, elle a donc supprimé l'article concerné. L'opération portant sur ADP a davantage divisé la commission spéciale. Si le caractère stratégique de l'entreprise et le précédent de la privatisation des autoroutes invitent naturellement à la méfiance, il m'a semblé néanmoins préférable de remédier aux lacunes du texte, de veiller à l'améliorer, plutôt que de s'y opposer frontalement et, sans doute, vainement. Dans cette optique, la commission spéciale a doté ce secteur du régulateur fort et indépendant qu'il mérite, tout en permettant aux collectivités territoriales de participer à l'appel d'offres de cession

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je voudrais vous dire dans quel état d'esprit la commission spéciale a abordé le chapitre III, « Des entreprises plus justes », et

de société européenne que nous entendons promouvoir. Enfin, ce texte contient également un certain nombre de demandes d'habilitation à légiférer par ordonnance. Je le dis clairement : la commission spéciale a souhaité restreindre autant que possible le recours aux ordonnances dans la mesure où nous considérons qu'il

Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission spéciale, madame, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, comme cela vient d'être exposé, le projet de loi comporte un ensemble de dispositions à caractère économique et financier. Ces matières sont très fortement marquées par le droit européen. Le marché intérieur est en effet largement harmonisé, même si les textes européens laissent des marges de manoeuvre aux États membres soit pour prévoir des mesures moins contraignantes, soit, au contraire, pour maintenir un droit national plus exigeant. La sur-transposition des textes européens en droit français porte atteinte, on le sait, à la compétitivité de notre économie. Dès lors, toute sur-transposition doit être identifiée, justifiée et proportionnée au regard d'objectifs d'intérêt général. C'est pour ce motif que la conférence des présidents a confié à la commission des affaires européennes, à titre expérimental, une mission d'alerte sur les sur-transpositions. Le projet de loi que nous examinons aujourd'hui constitue le quatrième exercice du genre, et je remercie de leur accueil la présidente et les rapporteurs de la commission spéciale. La commission des affaires européennes a constaté que le projet de loi supprime opportunément un certain nombre de sur-transpositions préexistantes, afin, en particulier, de renforcer l'attractivité de la place financière de Paris, à la veille du Brexit, qu'il s'agisse du relèvement du seuil de dispense de l'obligation d'établissement d'un prospectus en cas d'offre de titres au public, de l'abaissement du seuil de retrait obligatoire ou encore de la reconnaissance des systèmes de pays tiers pour le règlement définitif des opérations sur titres. Constitue également la suppression d'une sur-transposition le relèvement des seuils de contrôle légal des comptes des petites entreprises au niveau des seuils les plus élevés de la directive comptable- cela fait encore débat. Il s'inscrit dans l'objectif d'allégement des charges de ces entreprises. C'est aussi le cas de la publication simplifiée des comptes des moyennes entreprises, que le Sénat a étendue aux petites entreprises et aux micro-entreprises, leur permettant de ne plus être soumises à des obligations de transparence qui ne s'imposent pas à leurs concurrentes européennes. Il convient toutefois d'observer que ces mesures sont généralement « encadrées ». Soit parce qu'elles exploitent, mais dans certaines limites, des options ouvertes par les textes européens, soit parce qu'elles ajoutent une contrainte non prévue par ceux-ci. Tel est, par exemple, le cas des opérations dispensées de prospectus, pour lesquelles un document de présentation simplifié, déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers, devra être établi. Deuxième observation : le projet de loi renvoie très largement à des ordonnances pour la transposition de directives récentes- M. Canevet vient de s'exprimer à ce sujet -, au motif de la technicité des dispositions concernées et des coordinations à mettre en oeuvre. Cela se conçoit. Mais il conviendrait que l'habilitation indique précisément les options qui seront retenues. La commission spéciale a d'ailleurs souhaité procéder directement à la transposition dans la loi pour faire bénéficier les collectivités territoriales et leurs opérateurs du délai prorogé de mise en conformité autorisé par la directive sur la facturation dans le cadre des marchés publics. Ce cadrage initial est pourtant d'autant plus nécessaire que la ratification des ordonnances intervient souvent plusieurs mois, voire plusieurs années, après leur entrée en vigueur, ce qui ne permet pas au Parlement de revenir aisément sur les sur-transpositions qu'elles comportent. Je ne saurais conclure sans évoquer l'article 70 du projet de loi, qui modifie le régime comptable des grands ports maritimes pour tirer les conséquences d'une décision de la Commission européenne de juillet 2017. La question de la compétitivité des ports français et de l'appréhension de la spécificité de leurs activités au regard du droit européen ne saurait se limiter à cette seule disposition ! Nous passons

Vous l'avez maintes fois répété, ici même, dans de nombreux médias, car il serait, selon vous, urgent de libérer les entreprises. Mais le temps médiatique n'est pas le temps politique, et, vous en conviendrez, le buzz et la petite phrase ne font pas le débat politique. En près de dix ans, nous avons étudié six lois sur les entreprises, parfois sans attendre les effets de la précédente. Avec PACTE, nous sommes face à un mastodonte de près de 200 articles, qui s'attaque, pêle-mêle, aux seuils sociaux, à la Caisse des dépôts et consignations, à l'intéressement et la participation, et, enfin, aux privatisations. Au moins dix projets de loi en un seul, donc Nous regrettons le temps restreint pour discuter et auditionner en commission spéciale, d'autant que la procédure accélérée et la procédure de législation en commission pour certains articles ont raccourci nos débats. Oui, pour bien construire et voter une loi, il faut du temps. Et parfois, entre le dépôt et le vote à l'Assemblée nationale, puis ici au Sénat, les temps changent. un mouvement social s'est levé dans le pays, exigeant de la justice sociale, de la justice fiscale et une autre répartition des richesses. Pourquoi ne pas en parler, et peut-être légiférer sur une autre répartition des richesses créées par le travail, au chapitre III nous ne sommes pas seuls à voir que le climat social a changé. J'ai noté cette phrase : « L'idée que le prix de la croissance, ce sont les inégalités, est une idée injuste et une idée fausse. Nous ne pouvons pas payer toujours plus de croissance par toujours plus d'inégalités. Et si les responsables politiques, les chefs d'entreprise, les décideurs n'en prennent pas conscience, ce sont les peuples

dans un sens ni dans un autre sur la privatisation d'ADP ». Alors, essayons de dégager une majorité d'idées ! De quoi parlons-nous avec ADP ? Le groupe gère les 13 aéroports franciliens et détient des participations dans 26 aéroports de 30 pays différents. Ses revenus ont connu une augmentation annuelle moyenne de 3,8 %, et son résultat net a progressé de 10 %, depuis sa transformation en société anonyme. Alors que 102 millions de passagers ont utilisé les aéroports franciliens en 2017, Roissy-Charles-de-Gaulle devrait avoir à gérer un flux annuel millions de passagers d'ici à 2023, date de mise en service du terminal 4, ce qui en ferait le premier aéroport européen. qu'un aéroport est un bien commun et qu'il ne devrait pas avoir de valeur numéraire, à l'instar des gares, des ports, des autoroutes, des barrages hydrauliques, ou encore des monuments et sites historiques. Si élevé soit-il, le montant auquel la société aéroportuaire qui le gère sera vendue à des actionnaires privés ne pourra, selon nous, jamais compenser les coûts sociétaux et philosophiques du désengagement de l'État. Même les ultralibéraux disent : « Oui à la privatisation, mais dans le cadre d'une ouverture à la concurrence. » Un monopole naturel doit rester public. Le confier au privé revient à permettre à celui-ci de braquer la Banque de France en toute légalité et de faire fonctionner la machine à billets pour remplir les poches des actionnaires. Ce n'est pas acceptable Or nous avons des précédents. On pense évidemment aux privatisations des concessions autoroutières en 2006 : ces entreprises ont vu leurs actionnaires rentrer dans leur argent en moins de dix ans, tout en continuant à augmenter considérablement leurs profits en rackettant les automobilistes aux péages. En matière aéroportuaire, nous avons des exemples récents. En 2014, alors ministre de l'économie, Emmanuel Macron a bradé pour 308 millions d'euros les 49,9 % de parts de l'État dans la société de gestion de l'aéroport de Toulouse-Blagnac ... Eh oui ! ... à une entreprise chinoise, sans expérience dans la gestion des aéroports, domiciliée dans les îles Vierges britanniques et ayant une filiale dans les îles Caïmans, majoritairement contrôlée par l'État chinois. Il a confié à cet actionnaire privé l'entier contrôle de la société aéroportuaire toulousaine. Il y a une semaine, on apprenait que les Chinois voulaient revendre leurs parts pour 500 millions d'euros : jolie plus-value en cinq ans, pour des actionnaires rarement aperçus dans la cité rose, et qui n'ont pas investi un seul yuan pour développer l'aéroport. Et je ne parle pas des récidives, avec les aéroports de Nice et de Lyon. On nous dit Pas de panique, on a retenu la leçon. Cette fois-ci, on va bien négocier le cahier des charges. » Mais pour nous prononcer, monsieur le ministre, il faudrait encore que nous l'ayons sous les yeux, ce cahier des charges ! Exactement ! Ni les élus ni la direction ni les salariés ne l'ont vu, ne l'ont vu, et, comme le dit le vieil adage, « les promesses n'engagent que ceux qui les croient ». En réalité, nous assistons à un véritable démantèlement de la puissance publique et à la fin de l'État stratège.

et d'une stratégie globale, face à certains investisseurs étatiques étrangers. La définition d'un tel cadre par les instances récemment créées en matière de défense économique devrait être un préalable nécessaire à toute nouvelle cession d'actifs stratégiques. Est-il besoin de rappeler qu'ADP est la porte d'entrée sur notre territoire, notre vitrine pour le monde ? Qu'adviendra-t-il si, dans vingt ou trente ans, cette entreprise tombe entre les mains d'un investisseur étranger, comme celui de Toulouse-Blagnac, qui n'a pas les mêmes ambitions que nous pour notre territoire ? L'avenir de notre compagnie nationale, Air France, devrait d'ailleurs également nous préoccuper. Peut-on s'assurer que sa taxe aéroportuaire n'augmentera pas dans des mesures folles, ce qui mettrait à mal sa compétitivité ? Les Américains, eux, l'ont bien compris l'ensemble de leurs aéroports sont publics, notamment pour ne pas nuire à leur compagnie nationale. Nous ne sommes pas les seuls à être préoccupés. Les élus locaux, de leur côté, pointent deux questions. tout d'abord de la maîtrise du foncier, et donc de l'aménagement du territoire. ADP détient de nombreux terrains, notamment en Île-de-France, où s'exerce une forte pression foncière. On nous dit que le futur actionnaire ne pourra pas vendre sans autorisation de l'État ; nous aimerions plutôt que nos collectivités territoriales puissent être membres du conseil d'administration, sans devoir détenir des actions, pour être parties prenantes de l'aménagement du territoire. Il s'agit ensuite de l'impact social et des doutes quant à l'avenir des emplois, directs ou indirects, créés par ADP. Depuis l'ouverture du capital, 2 000 emplois ont été supprimés ; demain, qu'en sera-t-il, avec ADP à 100 % privé ? Monsieur le ministre, je ne peux pas ne pas évoquer votre principal argument, à savoir la création d'un fonds pour l'innovation. Vous attendez, de la vente des 50 % de parts que vous détenez, 8 à 10 milliards d'euros. Mais il faudra dédommager les actionnaires minoritaires, puisque leurs actions à vie vont devenir des actions à soixante-dix ans, ce qui aura un coût de 1 à 2 milliards

considérez-vous que 200 millions d'euros par an suffiront à concurrencer les Chinois et les Américains, notamment face aux défis que vous avez évoqués, comme le véhicule autonome, la robotisation de nos entreprises, la 5G ou l'intelligence artificielle

En tant qu'actionnaire minoritaire, détenant aujourd'hui 8 % des parts d'ADP, ce groupe sera indemnisé par l'État, en plus de l'indemnisation pour l'abandon de Notre-Dame-des-Landes. Il serait donc intéressant de savoir si c'est avec l'argent des contribuables qu'il va pouvoir racheter ADP J'ajoute qu'une question de constitutionnalité se pose avec l'alinéa 9 du préambule de 1946, repris dans le préambule de 1958 : « Tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a

je crois que personne n'a véritablement envie que les touristes atterrissant aujourd'hui à l'aéroport Paris-Roissy-Charles-de-Gaulle atterrissent demain à l'aéroport Paris-Roissy-Vinci car, plus qu'une infrastructure et un monopole naturel, c'est un peu de l'histoire de France que nous braderions ! Mes chers collègues, vous l'avez compris, nous nous opposerons à la privatisation d'ADP. J'espère que nous serons nombreuses et nombreux à mener ce combat ! La parole

présenté comme le grand texte économique de ce début de quinquennat, il se résume, pour l'essentiel, à diverses dispositions en matière économique, sans que les véritables enjeux soient traités de façon globale et cohérente. Sur la forme, le texte est passé de 73 articles à près de 200 à l'issue de son examen par l'Assemblée nationale. Au-delà de la diversité des sujets abordés et des mesures proposées, beaucoup de dispositions échappent donc à une étude d'impact, laquelle est pourtant obligatoire depuis 2008. Beaucoup de mesures échappent également au Parlement, puisque le nombre d'habilitations à légiférer par voie d'ordonnance, sur des sujets complexes parfois, était de quatorze quand le texte est arrivé sur le bureau du Sénat. y ait un véritable décalage entre les besoins des entreprises pour se développer, gagner des marchés et créer des emplois et les mesures contenues dans ce texte, dont on doute qu'elles permettent réellement de gagner en compétitivité. Par exemple, la définition de l'intérêt social et de la raison d'être de l'entreprise dans le code civil va indéniablement fragiliser les entreprises et faire peser sur elles un risque contentieux accru, alors que la législation française sur la responsabilité sociale La privatisation de monopoles, Aéroports de Paris et la Française des jeux, pour alimenter un fonds dont le rendement sera trop faible pour répondre aux enjeux, et alors même que d'autres dispositifs existent déjà, pose également question. Au total, il nous semble difficile de discerner une ligne directrice et d'estimer correctement quel sera l'effet de ce texte sur la croissance des entreprises. Et que dire de la cohérence de la politique économique du Gouvernement ? Les impôts de production, qui grèvent la compétitivité des entreprises, ne baissent pas. La France reste championne d'Europe en matière de prélèvements obligatoires et de dépenses publiques. Le déficit commercial se dégrade. Le ministre de l'économie prend souvent l'exemple du décrochage de la France par rapport à l'Allemagne. Mais, depuis quelques années, l'Allemagne a mis de l'ordre dans ses comptes publics- désormais, elle enregistre même des excédents budgétaires. Elle a taillé dans ses dépenses publiques, mis l'accent sur la compétitivité de ses entreprises, avec la baisse de la fiscalité et du coût du travail, avec une réforme des retraites, avec des efforts consacrés à l'apprentissage et à l'innovation. Le texte PACTE est loin de cette ambition. Pour autant, nous ne souhaitons pas que ce projet de loi soit rejeté en bloc. Des mesures vont indéniablement dans le bon sens et répondent aux attentes des entreprises la rationalisation des seuils, le délai de cinq ans pour répondre aux nouvelles obligations liées au franchissement d'un seuil, les dispositions pour développer l'intéressement et la participation, la mise en place d'un guichet unique pour la création d'entreprise et les démarches liées à son évolution, le mécanisme de liquidation judiciaire simplifiée, ou encore les mesures de simplification pour les micro-entrepreneurs et les créateurs d'entreprise. En outre, la commission spéciale a nettement amélioré le texte, notamment en allant plus loin sur la question des seuils, en assouplissant davantage le régime des actions de préférence, en abrogeant le droit d'information préalable des salariés en cas de cession de leur entreprise, qui peut compromettre les projets de reprise, en supprimant diverses sur-transpositions, en renforçant le cadre de régulation des crypto-actifs, en précisant le dispositif d'épargne retraite ou en harmonisant l'ensemble des taux dérogatoires du forfait social à 10 %. C'est ce travail-là que nous souhaitons poursuivre en séance publique. C'est pourquoi nous nous prononçons contre la motion tendant à opposer la question préalable, déposée par nos

dans l'objet de cette motion, vous indiquez que ce projet de loi est « un vaste chantier de dérégulation libérale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

Madame la présidente, monsieur le ministre, madame, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, nous commençons l'examen du projet de loi

transformer les entreprises françaises et les faire grandir ; simplifier et alléger la vie des entreprises ; et, enfin, donner un sens social à la vie en entreprise.

d'une désindustrialisation plus forte, qui se traduit par une offre de produits vieillissante et de qualité moyenne, d'une fiscalité trop lourde et mal répartie, et d'une structure d'entreprises déséquilibrée, que vous connaissez. La France dispose

par une vaste concertation. Dès le mois de novembre 2017, six groupes de travail associant des professionnels de différents domaines, des élus et des juristes se sont réunis et ont procédé à de nombreux travaux,

de la vie de l'entreprise ; la réforme de la profession de commissaire aux comptes ; la possibilité de rebond pour un professionnel, pour un entrepreneur, car, après tout, il n'est pas déshonorant d'échouer et l'on a le droit de recommencer, si c'est contraire à notre culture française ; la simplification des marchés financiers, des marchés participatifs, de l'assurance vie, de l'épargne retraite

dont on peut espérer qu'elle sera conclusive. Le PACTE est aussi un texte de justice sociale, avec la transparence des niveaux de rémunération

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi que nous avons à examiner est un véritable monstre législatif. Ce texte comportait initialement 71 articles, il en contient actuellement près de 200. Cette multitude d'articles aborde des sujets divers, en suivant une seule logique : favoriser le « business » à tout prix. Alors que les libertés fondamentales sont attaquées de toute part, seule la liberté d'entreprendre semble être au coeur des préoccupations du Gouvernement. Ce texte modifie le droit des sociétés, le droit financier et bancaire, le droit des entreprises en difficulté, des assurances, du travail, de la propriété intellectuelle et de la sécurité sociale. Chacun de ces thèmes aurait mérité un débat à part entière, tant les modifications sont importantes, d'un point de vue qualitatif comme quantitatif. Mais le choix du Gouvernement a été de raccourcir les débats pour aller vite. Comment accepter cette situation, alors que, dans la rue, nos concitoyens réclament davantage de démocratie ? Ces modifications sont divisées en trois parties : libérer les entreprises, les rendre plus innovantes et les rendre plus justes. Tout tourne donc autour de l'entreprise, ce qui conduit à s'interroger quant à sa place, quant au modèle de société que l'on veut promouvoir. Ce projet de loi prétend repenser la relation entre les entreprises et l'intérêt général. Mais il s'inscrit dans la continuité des précédentes réformes qui, additionnées les unes aux autres, conduisent à transformer profondément notre modèle social. Les reculs annoncés par cette loi sont nombreux : approfondissement du mouvement de financiarisation des entreprises, attaques contre nos mécanismes nationaux de solidarité et fragilisation des droits des salariés. Ainsi, après la loi El Khomri et les ordonnances Macron de septembre 2016, le projet de loi PACTE vient porter un nouveau coup aux droits des salariés. Derrière une volonté affichée et tant répétée la modification des seuils sociaux permet de revenir sur certaines obligations à la charge des entreprises, comme la mise à disposition d'un local syndical. Quant aux mesures censées favoriser la démocratie sociale, elles restent évidemment bien insuffisantes, tout comme le nombre de salariés présents dans les conseils d'administration et de surveillance, dont dont le pouvoir d'action est trop limité par le manque d'accès aux informations depuis la loi sur le secret des affaires. Nos systèmes de solidarité sont également Alors que le PLFSS pour 2019 a battu des records en matière d'exonération de cotisations sociales et que le principe de non-compensation par l'État a été acté, ce projet de loi continue de vider les caisses de la sécurité sociale. La modification des seuils sociaux et la suppression du forfait social représentent, à elles seules, un coût de 800 millions d'euros. Par ailleurs, plusieurs mesures annoncent la réforme à venir des retraites, à l'image des dispositions relatives à l'épargne salariale et des habilitations à réformer par ordonnances. Le Gouvernement entame donc la financiarisation de notre système de retraite, alors même que les concertations avec les syndicats sont encore en cours. Enfin, alors que ce projet de loi prétend vouloir repenser la place de l'entreprise dans la société, les mesures de dérégulation et de désengagement de l'État se multiplient. D'abord, le texte s'attaque aux chambres consulaires et aux chambres de métiers, malgré leurs missions de service public, essentielles à l'accompagnement des entreprises et à la formation professionnelle. Ensuite, et surtout, il procède à de multiples privatisations : la Française des jeux, Engie et Aéroports de Paris, dont mon collègue Fabien Gay vous a parlé. Le Gouvernement délaisse ainsi ses prérogatives d'État stratège et de régulateur. Après le fiasco de la vente des concessions autoroutières, il abandonne le secteur aérien à l'heure de la transition écologique, il livre Engie au marché et aux exigences de rentabilité à court terme. Quant à la vente de la Française des jeux, elle est tout simplement inquiétante quand on connaît les enjeux de santé publique. Le modèle social que nous défendons est complètement à l'opposé de celui qui nous est proposé ici et qui repose sur la fragilisation du droit du travail, sur l'attaque contre les services publics et les systèmes de solidarité, sur le désengagement de l'État et sur la dérégulation des marchés financiers. Ce projet de loi s'appuie sur des présupposés idéologiques et économiques mis en oeuvre depuis des décennies, qui n'ont pas démontré leurs effets en matière de pouvoir d'achat et de justice sociale et qui fragilisent les salariés. Nous nous opposons au mouvement de financiarisation de l'entreprise et de la société en général, qui est au coeur de ce texte. Pour rappel, selon l'INSEE, de 1980 à 2015, la part des dividendes est passée de 3 % de la richesse nationale à 10 % en euros constants. Cette financiarisation des entreprises empêche de prendre en compte l'ensemble des enjeux sociétaux, comme l'environnement, la démocratie sociale ou la collectivité dans laquelle l'entreprise est insérée. C'est pourquoi la finalité de l'entreprise ne doit plus être la production de biens et de services et la rentabilité à court terme. Parce que ce projet de loi est complètement à l'opposé de ce que nous défendons, nous voterons contre !

Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission spéciale, madame, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, lorsqu'un gouvernement a l'ambition de « relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, pour renouer avec l'esprit de conquête économique », on ne peut que saluer cette volonté. On se dit même que l'on va enfin pouvoir débattre de la place de l'entreprise française dans l'économie nationale et mondiale. Force est de constater que ce texte arrive très tard, vous l'avez dit vous-même, monsieur le ministre. On peut imaginer que, il y a quelques mois, il vous aurait permis d'acquérir, par exemple, des outils pour contrer plus tôt la décision de Ford à Blanquefort. Aujourd'hui, il arrive finalement presque trop tôt, puisqu'il ne permettra pas de prendre en compte les propositions qui émergeront du débat national qui commence. Monsieur le ministre, vous avez indiqué hier que vous souhaitiez « construire un capitalisme nouveau, capable de lutter contre les inégalités, et mettre fin à des excès qui ont compromis son succès et son efficacité.

que dans celui du « renouer », du « défaire » plutôt que du « faire », du « démantèlement » plutôt que de la vision d'un État stratège. Selon nous, un système économique ne peut s'affranchir de la justice sociale, ni même d'une équitable répartition des richesses entre le patron, l'ouvrier et la puissance publique. L'État a un rôle à jouer en donnant les outils nécessaires pour que les entrepreneurs se sentent libres et en sécurité de créer et/ou d'investir dans une TPE-PME et que les salariés obtiennent une juste reconnaissance de leur activité, par le biais d'un salaire décent ou d'une association à la prise de décision.

quel projet économique voulons-nous pour notre société demain ? Quel lien dresser entre la société et l'appareil productif ? Comment est associée et valorisée la force de production du salarié dans le cadre de ce développement économique ? Quels outils de développement économique apporter à l'économie de proximité ? Aujourd'hui, le débat s'attache principalement à la financiarisation des entreprises plutôt qu'à leur capacité d'innovation et d'investissement, comme il y a maintenant trente ans. Nous considérons pourtant que c'est cette dernière qui permet de créer de la valeur économique.

Les grandes entreprises sont considérées, quand les tissus économiques locaux et régionaux de notre pays sont abîmés. La pérennité de l'État stratège est mise à mal. Que devient notre rôle dans la fixation du cap économique à donner à la France ? Les obligations des entreprises, très souvent appelées, sans doute parfois à tort, « contraintes », sont largement allégées, alors que la prise en compte du salarié est timidement accrue. Je voudrais revenir sur certaines dispositions du texte qui témoignent du sophisme induit par un terme que vous utilisez souvent : « liberté ». Est-ce redonner de la liberté aux entrepreneurs que de leur supprimer le stage de préparation à l'installation, lorsque l'on sait que, si la France crée beaucoup d'entreprises, peu nombreuses sont celles qui passent le cap de la première année d'existence ? Est-ce aider nos TPE et nos PME que de vider les CCI de leur mission de service public plutôt que de leur suggérer des plans de restructuration et des outils de développement en matière d'export, peut-être avec le concours de Business France et de Bpifrance ? Pensez-vous que, au regard de l'actualité et de la demande urgente de formation, d'accompagnement et d'emploi au plus près des territoires que les citoyens ont exprimée, il soit pertinent de mutualiser les moyens accordés aux CCI, dont on sait que les premières à disparaître seront celles des territoires ruraux ?

correspond non pas à la définition de « libérer », mais plutôt à celle de « libéraliser », ce qui revient à demander aux Françaises et aux Français qui souhaitent devenir entrepreneurs de construire une maison sans outils ni matériaux. Le projet de loi PACTE passe à côté de l'objectif affiché de mieux partager la valeur dans les entreprises. Au-delà de l'épargne salariale, les vrais enjeux résident dans les écarts de rémunération, dans le partage entre dividendes et salaires ainsi que dans la participation des salariés à la vie et aux décisions de l'entreprise. sont pourtant totalement oubliés du texte gouvernemental. À l'heure où le mouvement des « gilets jaunes » a rappelé au Gouvernement les attentes des Français en matière de justice sociale et de lutte contre les inégalités, nous regrettons l'absence de propositions du Gouvernement sur ces questions.

C'est ainsi seulement que l'on repensera véritablement leur place dans la société. Nous proposons une vraie implication des salariés dans la vie et dans la gestion des entreprises. En outre, nous entendons protéger les entreprises contre les dérives de la financiarisation de l'économie, en faisant primer l'emploi et le long terme sur le cours de la bourse, en leur interdisant de s'endetter pour verser des dividendes aux actionnaires-

La privatisation d'entreprises stratégiques et rentables, telles qu'Engie, la Française des jeux et Aéroports de Paris, ainsi que leur alignement sur le modèle privé, se fera au détriment des recettes de l'État, affaiblira le service public

le secteur public n'est pas moins performant que le secteur privé, bien au contraire. Vous devez ainsi garder en main les outils de structuration de la politique économique et, plus encore, renforcer des filières stratégiques, qui sont la garantie de l'indépendance de notre pays.

au sens constitutionnel ; il serait donc souhaitable qu'elle demeure une propriété de la collectivité. En outre, elle a rapporté 258 millions d'euros de dividendes en 2016 au budget de l'État. Brader ADP reviendrait donc à sacrifier notre politique d'aménagement du territoire et des mobilités sur l'autel d'un fonds de liquidités qui sera écoulé en

Cela mettrait également la France dans une situation inédite : en Europe comme dans le reste du monde, à l'exception de l'Australie, les États sont au capital de leurs sociétés d'aéroports, sans doute parce qu'ils y voient un intérêt économique, politique et stratégique. Sommes-nous plus visionnaires que les autres ? En aucun cas ! La situation de l'aéroport de Toulouse ne vous aura pas échappé et le rapport de la Cour des comptes qui « tacle » sa privatisation devrait, plus que jamais, vous alerter : pas d'investissements, contrairement à ce qui avait été promis, pillage des réserves et, maintenant, une vente en perspective, avec une plus-value de 192 millions d'euros pour le consortium chinois acquéreur. Voilà un bel exemple de spéculation financière sur des outils de mobilité stratégiques pour notre pays

Plus loin, le même ajoute : « Celles et ceux, que j'ai pu entendre, qui s'indignent de cette cession minoritaire de la société de gestion de l'aéroport de Toulouse ont pour profession, d'une part, d'invectiver le Gouvernement et, d'autre part, d'inquiéter les Français. » Non, monsieur le ministre, nous ne sommes pas là pour inquiéter les Français, nous entendons défendre leurs intérêts.

Enfin, concernant la privatisation d'Engie, outre le risque de recul en matière de sécurité de l'approvisionnement énergétique de la France, une telle orientation se traduira par un renchérissement probable du prix de l'électricité et du gaz pour nos concitoyens.

s'il s'agit incontestablement d'un texte intéressant, dont on ne peut qu'approuver les orientations générales, il contient cependant des dispositions assez disparates, allant de la suppression du stage à l'installation des artisans à la privatisation de trois grands groupes publics, en passant par la possibilité de définir une « raison d'être » de l'entreprise. Je qualifierais plutôt ce texte d'étape importante dans l'adaptation à la transformation de notre économie. place des conditions favorables à la création et au développement des entreprises et essaie de mieux associer les salariés à cette démarche. La simplification, la réduction des délais, l'allégement des contraintes et la dématérialisation y sont très souvent mis en avant. Attention, toutefois : entre les mots et la réalité concrète de la vie de l'entreprise, il y a parfois des écarts qui, lorsqu'ils sont trop flagrants, peuvent provoquer des frustrations et des déceptions. que la complexification coure plus vite que la simplification ! Sauf à faire un examen exhaustif des différentes mesures, je vais rapidement évoquer celles qui me paraissent les plus satisfaisantes, celles qui mériteraient d'être améliorées ou enrichies et celles, enfin, qui ne nous ont pas convaincus.

une PME de mon département qui a fait l'objet d'une transmission familiale. Le fondateur, qui est toujours le principal actionnaire, se trouvait dans l'entreprise et apportait son concours à son fils dans différentes tâches.

; augmentation du nombre d'administrateurs salariés dans les conseils d'administration ou de surveillance ; réforme de l'épargne, avec notamment la promotion du PEA-PME et un meilleur fléchage de l'assurance vie en direction de l'actionnariat, donc des entreprises ; protection des entreprises stratégiques, avec le renforcement de la procédure d'autorisation préalable d'investissement. Il y a, enfin, la suppression du forfait social sur l'intéressement pour les entreprises de moins de 250 salariés et sur la participation pour les entreprises de moins de 50 salariés. Sur ce dernier point, monsieur le ministre, je vous ferai une proposition, ainsi que nous en avons déjà parlé, consistant à étendre le champ d'application obligatoire de l'intéressement à toutes les entreprises à partir de 11 salariés, dès lors qu'elles n'ont pas institué de participation. C'est dans l'intérêt des entreprises, en termes de motivation du personnel, comme dans celui des salariés, dans l'optique d'une meilleure répartition des richesses et d'une amélioration du pouvoir d'achat. Dans le contexte actuel, cette disposition ne pourrait que contribuer à crédibiliser la démarche du Gouvernement dans le cadre du grand débat national. Parmi les sujets qui soulèvent certaines difficultés, il y a, bien entendu, la restructuration des réseaux consulaires. Si nous sommes favorables à des contraintes de mutualisation, nous ne sommes pas pour autant convaincus par la régionalisation des chambres de métiers, qui se traduira nécessairement, à terme, par une nouvelle perte de proximité pour les structures départementales. Par ailleurs, le stage d'accompagnement à l'installation, à condition de le cibler strictement sur les aspects relatifs à la gestion, mérite d'être maintenu pour les candidats n'ayant aucune notion dans ce domaine ; les autres en sont déjà exonérés. Sa suppression offre, certes, un affichage de simplification, mais elle ne rendrait pas service aux artisans. Je m'interroge également sur l'absence dans ce texte de propositions d'amélioration significative du droit des sociétés ou encore de solutions aux freins existants pour les entreprises dans l'accès au crédit, qui n'est traité que par le biais de la commande publique- de manière positive, d'ailleurs -et de l'orientation des capitaux, ce qui, en pratique, ne répond pas totalement aux besoins exprimés par les PME pour financer leurs investissements et leur fonds de roulement. Le secteur bancaire, qui n'est pratiquement pas évoqué en dehors de la Caisse des dépôts et de La Poste, demeure extrêmement frileux nous interrogeons également sur les conditions de privatisation de trois grands groupes et sur le contrôle que l'État doit conserver sur la mise en oeuvre des missions dont ceux-ci ont la charge. Si la destination de ces cessions de participations publiques permet la constitution d'un fonds pour l'innovation et l'industrie- une excellente utilisation on ne peut cependant réprimer certaines craintes au vu des expériences passées, comme celle des sociétés d'autoroutes ou encore de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, au sujet desquelles on a bien constaté que les plus-values potentielles d'exploitation étaient plus facilement captées par les opérateurs privés, bien meilleurs que l'État

En conclusion, le groupe du RDSE émettra un avis très majoritairement favorable sur ce texte, en espérant que des améliorations puissent intervenir au cours de l'examen que nous engageons ce jour.

Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission spéciale, madame, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, je souhaite en premier lieu remercier le Gouvernement d'avoir mis ce texte à l'ordre du jour. Il m'arrive parfois d'être assez critique, mais il n'y a pas de raison de l'être systématiquement ! Bien sûr, on peut regretter que ce texte contienne des propositions assez disparates qui nuisent à la cohérence de l'ensemble on peut regretter que la privatisation d'ADP ou de la Française des jeux n'ait pas fait l'objet d'un texte séparé ; mais nous devons nous réjouir de l'occasion qui nous est donnée de pouvoir enfin légiférer sur les effets de seuil et autres simplifications administratives.

ce seul point ! J'en profite pour souligner la qualité du travail accompli par la commission spéciale sous votre autorité, madame la présidente, ainsi que le travail précis des rapporteurs et de l'administration du Sénat.

il me paraît indispensable que l'État reste majoritaire dans ADP, ou, en tout état de cause, qu'il conserve une capacité d'intervention très forte. Les privatisations doivent être envisagées sous l'angle d'un meilleur fonctionnement ou d'un désendettement, sinon elles ne sont que des remèdes à court terme. J'ai bien entendu vos explications, monsieur le ministre. Elles me montrent que je n'ai peut-être pas fait le tour de la question et que celle-ci mérite d'y réfléchir encore.

monsieur le ministre, madame la présidente de la commission spéciale, madame, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues,

Le Gouvernement a fait le choix d'une procédure accélérée pour l'examen de ce projet. Cette décision, toujours dommageable pour la qualité de nos débats, répond à l'impatience de nos concitoyens de voir levés nombre des obstacles qui brident leur volonté d'entreprendre. Le Gouvernement, qui avait annoncé l'élaboration du projet de loi dès les premiers mois du quinquennat, a aussi fait le choix de consulter assez largement en amont pour coconstruire le texte avec la société civile, afin de dresser un diagnostic aussi complet que possible de ces obstacles et d'y apporter des réponses pragmatiques. Cette méthode ne me semble pas la moins bien adaptée face à l'ampleur de l'enjeu. cependant aussi ses inconvénients : le texte contient de très nombreuses mesures, au risque de l'éparpillement, voire, parfois, de la confusion. Le groupe Les Indépendants veillera autant que faire se peut à ce que le projet conserve une cohérence conforme à son ambition initiale : faire grandir les entreprises et mieux partager la valeur. Ce texte va très clairement dans le bon sens. En levant les freins à la création d'entreprise, il favorise la liberté d'entreprendre qui se trouve au fondement de nos valeurs. Nous soutiendrons donc les mesures qui facilitent la prise d'initiative, comme la simplification et l'harmonisation des seuils d'effectifs ou la création du guichet unique pour les entrepreneurs. Lever ces freins à l'initiative individuelle contribuera à rendre notre économie plus inclusive, mais cela ne suffira pas : il faut également travailler à aligner les intérêts des salariés sur ceux de l'entreprise. C'est pourquoi nous soutiendrons également la suppression partielle partielle du forfait social sur la participation et l'intéressement. Nous proposons même d'aller plus loin, en étendant cette mesure aux ETI qui concluent des accords de participation au-delà de leur obligation légale. Cela emporterait des effets concrets pour les PME et les ETI qui investissent et créent des emplois au coeur de nos territoires. Pour changer la place de l'entreprise dans notre société, nous croyons davantage à ce type de mesures concrètes et pragmatiques qu'aux grandes déclarations de principes. nous ne vous cachons pas notre réserve à l'égard de la modification de l'objet social de l'entreprise, qui risque de constituer une atteinte à la liberté d'entreprendre et, surtout, une source d'insécurité juridique permanente. Mes chers collègues, gardons à l'esprit un principe : la transformation de notre économie ne se décrète pas, elle échoit aux entreprises qui se développent. Tâchons de mettre à leur disposition les bons outils pour accélérer leur croissance. C'est ainsi qu'elles continueront d'investir et d'innover pour se transformer et s'adapter aux évolutions de l'économie, c'est ainsi qu'elles inventeront un nouveau modèle d'entreprise qui façonnera l'avenir d'un capitalisme plus humain. Un chapitre entier du projet de loi est consacré aux entreprises plus innovantes ; en son sein, un volet important porte sur la seule question du financement. Dans ce domaine aussi, des actions très concrètes devraient permettre de rendre notre environnement réglementaire plus attractif pour les entrepreneurs qui innovent en France. Le Gouvernement a d'ailleurs fait le choix de se désengager du capital de certaines entreprises pour contribuer au financement de l'innovation. Je ne partage pas un certain nombre de critiques

À cet égard, monsieur le ministre, je partage votre opinion selon laquelle les boutiques de luxe des aéroports n'ont pas à être gérées par l'État, dont ce n'est pas le métier.

Bien sûr, ce projet de loi ne résoudra pas tous les problèmes, loin s'en faut, et le Gouvernement devra poursuivre l'effort engagé pour réduire les prélèvements obligatoires sur les entreprises, ce qui suppose de poursuivre également l'effort engagé pour réduire les dépenses publiques. Le groupe Les Indépendants n'en salue pas moins la volonté du Gouvernement d'alléger les contraintes qui pèsent sur nos entreprises. Nous soutiendrons donc les dispositions qui leur permettront de créer plus de richesses et de mieux les partager. Elles redonneront à nos entreprises des marges de manoeuvre pour continuer à investir et à créer de l'emploi en France. Tel doit être notre seul cap en matière de politique économique

Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission spéciale, madame, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, si ce « PACTE » est pavé de bonnes intentions, nous regrettons de devoir l'examiner en procédure accélérée. Il ne faut jamais confondre vitesse et précipitation ... À l'examen de ce texte, la première impression pourrait être bonne, toute une série de mesures semblent aller dans le bon sens et répondre aux attentes des entreprises : la rationalisation des seuils, le délai de cinq ans pour répondre aux nouvelles obligations liées au franchissement d'un seuil, les dispositions pour développer l'intéressement et la participation, la mise en place d'un guichet unique pour la création d'une entreprise et les démarches liées à l'évolution de celle-ci, le mécanisme de liquidation judiciaire simplifiée et les mesures de simplification pour les micro-entrepreneurs et les créateurs d'entreprise. Malheureusement, à y regarder de plus près, il semble qu'il y ait un véritable décalage entre les besoins des entreprises pour se développer, gagner des marchés et créer des emplois et les mesures contenues dans ce texte, dont on doute qu'elles permettent réellement de gagner en compétitivité. Les bonnes intentions sont là, mais la complexité administrative est toujours un frein à la compétitivité des entreprises françaises. Certaines dispositions du texte ne vont pas assez loin, notamment en matière de simplification. Nous ferons plusieurs propositions complémentaires au cours des débats, la diminution du volume normatif pour les entreprises, l'entrée en vigueur groupée des nouvelles règles s'imposant aux entreprises et la déclaration fiscale unique. D'autres dispositions demandent une vigilance accrue. C'est le cas, notamment, de la définition de l'intérêt social et de la raison d'être de l'entreprise dans le code civil, qui ne doit pas se transformer en une contrainte supplémentaire. Nous proposerons de supprimer cette disposition, qui fait peser sur les entreprises un risque contentieux accru. C'est le cas, également, du fonds pour l'innovation et l'industrie, qui nécessiterait les privatisations voulues par le Gouvernement pour l'alimenter. Pourquoi céder des monopoles publics rentables et stratégiques, alors que les dividendes actuels de ces sociétés, sans effort ni ambition particulière de la part de l'État, correspondent aux rendements annuels attendus du fonds ? avec lui, d'un aéroport-capitale, aéroport-frontière, engendrerait des déséquilibres dans les territoires, un risque de spéculation foncière et des conséquences économiques pour les compagnies aériennes, avec un risque de fluctuation

Nous sommes las des projets de loi du « en même temps ». Votre volonté de simplification du monde de l'entreprise est l'arbre qui cache la forêt d'autres décisions déterminantes, qui s'avéreraient, à terme, préjudiciables à l'avenir de notre pays.

libérer les énergies, c'est aussi libérer la possibilité pour les représentants des territoires de s'organiser comme ils le souhaitent, en responsabilité ! Pour aménager la régionalisation prévue par le texte, je proposerai donc un amendement de réécriture de l'article 13 A, visant à ne pas vider de leur substance des entités qui fonctionnent bien et qui refusent de se voir imposer un centralisme régional, au détriment de l'action de proximité sur les territoires départementaux. s'assurer une légitimité et une lisibilité, ainsi qu'un pouvoir d'action, en plus de réels moyens, est primordial pour les chambres départementales de métiers et de l'artisanat. et de l'artisanat. Par-dessus tout, avec ce projet de loi, c'est la question de la cohérence de la politique du Gouvernement en matière économique qui se pose les impôts de production, qui grèvent la compétitivité des entreprises françaises, ne baissent pas, la France reste championne d'Europe en matière de prélèvements obligatoires et de dépenses publiques, et le déficit commercial se dégrade. Monsieur le ministre, vous mentionnez souvent le décrochage de la France par rapport à l'Allemagne. Mais l'Allemagne a, depuis quelques années, mis de l'ordre dans ses comptes publics, enregistrant même des excédents budgétaires,

Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission spéciale, madame, messieurs les rapporteurs, le projet de loi PACTE, qui est un véritable enjeu, déclenche un certain nombre de passions, et plutôt de postures. Aujourd'hui, je voudrais rappeler quel est le défi

En même temps, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut favoriser l'emploi. Il faut favoriser l'emploi, mais, comme certains ne veulent plus trop de chefs d'entreprise, il faut bien sûr favoriser l'initiative personnelle. Très bien ! C'est d'une certaine

le ministre, est en votre faveur : vous avez pris le temps d'écouter, de consulter et de travailler avec les chefs d'entreprise et les représentants syndicaux pour essayer de faire ressortir un certain nombre de priorités.

monsieur le ministre, réduire à tout prix n'est pas forcément un objectif. Se pose aussi le problème de l'accompagnement d'un certain nombre de créateurs d'entreprise. Tout le monde connaît le rôle important d'appui à la création joué par les chambres consulaires, notamment les chambres de métiers. Je pense véritablement qu'on ne des personnes, des jeunes, dans une création d'entreprise sans leur apporter un minimum d'appui et de formation au départ, mais aussi d'accompagnement dans le temps. Les entreprises qui réussissent sont celles qui sont accompagnées durablement

ruraux ? N'est-on pas capable de laisser à l'initiative des chambres consulaires leur organisation régionale, peut-être sur le plan administratif, leur occupation du territoire et leur présence sur le terrain,

un projet de loi visant l'amélioration de la vie des entreprises. On l'attendait avec impatience, pensant qu'un certain nombre de mesures révolutionneraient le monde des entreprises.

qui n'est pas en mesure de défendre correctement ses intérêts. À ce stade de la procédure budgétaire, je tiens à remercier la présidente de la commission spéciale et le rapporteur chargé du volet « privatisations » de nous permettre d'avoir un débat public.

quatorze ans, sous Jacques Chirac, l'établissement public a été transformé en société anonyme. Puis le capital a été ouvert, en 2006, par une mise en bourse. En novembre 2008, sous Nicolas Sarkozy, le groupe Schiphol est entré au capital d'ADP.

Il y a des aéroports publics bien gérés et d'autres qui le sont moins ; il en est de même dans le secteur privé. La question me paraît être : dans quel cadre les aéroports opèrent-ils, et les intérêts de l'État et du transport aérien sont-ils bien garantis S'agissant des intérêts de l'État, le risque serait, comme il a été indiqué, de reproduire ce qui s'est passé pour les autoroutes. Ce risque me paraît devoir être écarté, au vu des dispositions adoptées par l'Assemblée nationale. M. le ministre en parlé, et je pense qu'il pourra être encore plus loquace sur le sujet.

Deux questions viennent ensuite. D'abord, est-ce le rôle de l'État d'être actionnaire d'aéroports, alors qu'il garde le contrôle aérien, la gestion des droits de trafic, la police aux frontières, la douane et la sécurité ?

que les compagnies souhaitent un régulateur indépendant, qui les préserve des augmentations de redevances. Ce n'est pas que la cession d'ADP les enthousiasme, mais elles soulignent que celle-ci ne doit pas être opérée à leur détriment et nous invitent à amender le texte dans le sens d'un renforcement

Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission spéciale, madame, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, un plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, soit

Le premier élément à relever, c'est que quasiment aucune obligation nouvelle ni contrainte supplémentaire n'est inventée pour les entreprises. C'est suffisamment rare pour être souligné ! La simplification des seuils sociaux est également une véritable avancée. La multiplicité de ces fameux seuils constituait un réel frein au développement des entreprises. En revanche, avec le seuil de 50 salariés, n'est-on pas dans la demi-mesure ? En effet, on peut légitimement être inquiet pour les PME de plus de 50 personnes, celles, précisément, qui sont le maillon faible de l'économie française.

Cette mesure devrait inciter à associer davantage les salariés aux résultats de l'entreprise, ce qui est une bonne chose. Mais chassez le naturel, il revient au galop : derrière de bonnes intentions, on nous refait le coup de la loi fourre-tout Nous avons tous en mémoire l'ineffable loi pour un État au service d'une société de confiance, espèce de baudruche administrative accouchant d'une souris Pas plus qu'il n'est possible de réformer l'administration en utilisant les outils qui, précisément, rendent l'administration française lourde, coûteuse et bureaucratique, il n'est possible de transformer le monde de l'entreprise, quels que soient les instruments juridiques dont on dispose et que l'on doit mettre en oeuvre, sans un vrai changement de culture. La modification de la notion d'objet social doit-elle être comprise comme cela ? Si c'est le cas, c'est un peu court, car la jurisprudence risque, demain, de transformer une bonne intention en épée de Damoclès redoutable pesant sur la tête de nos entreprises.

Rendez-vous compte : les mêmes qui, hier, ont bradé scandaleusement les autoroutes et ont le culot de soutenir, aujourd'hui encore, que l'État a fait une bonne affaire, sont prêts à nous refaire le coup, cette fois avec Aéroports de Paris. On en est réduit à liquider les bijoux de famille, ni plus ni moins : on continue à vider la baignoire, sans arrêter le robinet. Il faut se pincer pour y croire Bien sûr, nous en débattrons dans cet hémicycle : c'est une excellente chose, car, jusqu'à plus ample informé, la démocratie fonctionne ainsi. Dans le climat social désastreux que traverse notre pays, chacun prendra ses responsabilités. Monsieur le ministre, parallèlement au débat parlementaire, pourquoi ne pas suggérer à vos collègues Sébastien Lecornu et Emmanuelle Wargon de poser la question de la privatisation d'ADP dans le cadre du grand débat national ? Je vous garantis le résultat ne nous y trompons pas : pour libérer nos entreprises, il y a loin de la coupe aux lèvres avec ce « PACTE ». Rien dans ce texte sur la transition numérique, qui conditionne pourtant l'avenir de nos entreprises. Rien non plus pour favoriser les transmissions d'entreprise, alors que l'on sait pertinemment que plus de 500 000 entreprises seront à reprendre dans les dix prochaines années. Alors oui, alléger les contraintes est la voie à emprunter pour redynamiser notre tissu économique et montrer enfin à ceux qui entreprennent que la Nation est derrière eux. Mais faisons-le réellement

texte : permettre à nos entreprises de grandir, de se développer, de se créer et d'investir plus librement ; supprimer un certain nombre de contraintes. Comme cela vient d'être rappelé, ce texte ne comporte aucune nouvelle obligation pour les entreprises.

plus de taxe sur l'intéressement pour tous les salariés des entreprises de moins de 250 salariés. C'est une évolution en profondeur, ce n'est pas une « pichenette » ! C'est la sécu qui paie ? C'est une transformation majeure. Vous auriez également pu évoquer- personne n'en a parlé -, la transformation de l'épargne salariale, car cela concerne la vie quotidienne des salariés.

J'entends, sur les travées de gauche, des récriminations sur ce sujet, mais, enfin, vous devriez être révoltés de voir que notre pays est aujourd'hui, en Europe, celui qui conserve le taux de chômage le plus élevé, parce que nous n'avons pas eu le courage de libérer la capacité d'embauche de nos entreprises, de nos PME, des commerçants, des artisans, de tous ceux qui créent des emplois dans le pays vous pouvez garder les mêmes vieilles recettes qui ont échoué depuis trente ans et qui expliquent la crise dans laquelle nous sommes aujourd'hui, ou vous pouvez essayer de changer de direction, et c'est ce que nous proposons avec le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises. Oui, nos entreprises ont besoin de capitaux. Oui, elles ont besoin de financer. Oui, elles ont besoin d'investissements. Mais tant que l'on mentira aux Français sur la nécessité pour les entreprises d'avoir plus de liberté,

comptent parmi les plus pauvres et les plus démunis de la société française. Il est temps d'essayer autre chose, et c'est ce que nous faisons avec ce projet de loi ! J'en viens aux privatisations. Libre à vous d'estimer que, en matière d'innovation,

pour investir dans ADP, nous préférons financer l'investissement, l'innovation et la souveraineté technologique de la France. que ces choix fondamentaux, qui sous-tendent le projet de loi PACTE, permettront aux entreprises de grandir. Mieux rémunérer et associer les salariés, redéfinir la place respective de l'État et de l'entreprise dans la nation française, c'est une voie nouvelle qui doit nous permettre de remédier aux échecs français depuis trente ans : le chômage de masse, la lourdeur administrative, les contraintes pesant sur les entreprises, la mauvaise association des salariés et l'insuffisante rémunération des salariés pour le travail qu'ils accomplissent, le bridage des capacités d'investissement, d'innovation, de recherche et de créativité propres au peuple français.

Si des voyageurs veulent passer par un autre aéroport que celui de Roissy-Charles-de-Gaulle, ils peuvent parfaitement le faire et s'affranchir, avec la liberté la plus totale, de passer par Paris pour leurs vols longs courriers ; c'est d'ailleurs ce qui se passe dans bien des cas lorsqu'un

de ne pas jouer avec les peurs des Français concernant le contrôle de l'État ou la capacité que nous avons à protéger nos frontières. Le contrôle aérien, comme cela a d'ailleurs été rappelé précédemment avec beaucoup de justesse, reste aux mains de l'État. La gestion des trafics

Je crois profondément que nous avons besoin de passer à autre chose en matière économique. Il nous faut transformer en profondeur notre économie pour qu'elle crée plus de prospérité, plus d'emplois et qu'elle permette au génie français de s'exprimer avec toute l'ampleur dont il est capable. Ce n'était

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, mon rappel au règlement se fonde sur l'article 45 de la Constitution : « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien direct, même indirect, avec le texte déposé ou transmis

cet article. L'accompagnement psychologique des entrepreneurs dont l'entreprise connaît des difficultés n'a-t-il pas un lien direct avec le rebond des entreprises ? amendements relatifs à l'allotissement et à la commande publique n'ont-ils pas un rapport avec le rebond et la santé des entreprises quand on sait que trois directives européennes nous obligent à allotir et faire en sorte que- enfin

d'euros étaient redonnés aux familles, rien que pour cette assurance. Des sociétés de courtage et d'assurance ont trouvé un développement extraordinaire. Cela n'a-t-il pas un lien avec la santé des entreprises ? Aussi, l'article 45 a été appliqué d'une façon parfois contradictoire, mais surtout restrictive.

72, 73 et 74 -de ce projet de loi font l'objet d'une procédure de législation en commission. Le vote sur l'ensemble de ces articles est donc réservé jusqu'avant le vote sur l'ensemble du texte.

mes chers collègues, avant que ne s'engage la discussion des articles, permettez-moi de dire quelques mots en tant que présidente de cette commission spéciale. Tout d'abord, je veux remercier de leur travail nos trois rapporteurs, les administrateurs, ainsi que l'ensemble des membres de la commission spéciale pour leur participation. Nos débats furent parfois vifs, dans le respect de chacun toutefois, animés par nos convictions diverses, mais toujours avec la même préoccupation, celle d'apporter au texte une valeur ajoutée. Je suis sûre que les débats en séance publique se dérouleront dans le même esprit. Je souhaite insister sur le temps que nous avons consacré à l'écoute de tous ceux qui sont concernés directement ou indirectement par les dispositions du projet de loi. Je sais que certains membres de la commission spéciale ont regretté les conditions du débat parlementaire- trop peu de temps ; trop de sujets abordés, qui auraient souvent demandé à être traités spécifiquement et non pas dans l'urgence mais je dois rappeler que nous avons reçu, dans le cadre des auditions ouvertes à tous les membres de la commission spéciale, plus de 320 personnes et de très nombreuses contributions écrites. Néanmoins, je voudrais vous faire part de mon étonnement vous concernant, monsieur le ministre.

comme décourageants, parfois affligeants et particulièrement offensants pour la chambre haute. Comment pouvez-vous affirmer que ce sont les chambres parlementaires, et plus précisément le Sénat, qui empêchent les entreprises de se développer et la croissance de repartir, sous prétexte que la procédure législative serait insupportablement lente et provoquerait le blocage de votre projet de loi Faut-il vous rappeler que c'est vous qui avez entamé en amont une longue concertation avec les entreprises et les différents syndicats, que c'est vous qui avez déposé, le 19 juin 2018, le texte devant l'Assemblée nationale, et ce en procédure accélérée Adopté le 9 octobre 2018 par l'Assemblée nationale, le texte est arrivé sur le bureau du Sénat le 10 octobre 2018, avec 123 articles supplémentaires. Vous êtes, avec le Gouvernement, le chef d'orchestre de l'inscription des textes au calendrier parlementaire. Où y voyez-vous notre lenteur parlementaire ? La commission spéciale que j'ai l'honneur de présider a consacré onze semaines et demie à l'examen d'un texte comprenant 196 articles ; cela me semble raisonnable lorsque l'on sait que seuls 73 articles ont fait l'objet d'une étude d'impact. vous constaterez tout l'intérêt d'une seconde chambre pour simplifier et enrichir ce texte, comme vous l'avez d'ailleurs vous-même dit il y a un instant. Le Parlement n'est pas là pour ralentir, mais bien pour améliorer.

Madame la présidente, nous n'avons pas dû écouter la même émission. Je ne me serais jamais permis,

En revanche, ceux qui me connaissent ici savent que je défends depuis des années, avec beaucoup de constance, une refonte du système politique français et de nos procédures. Ce n'est pas le Sénat, l'Assemblée nationale, l'exécutif ou le fonctionnement gouvernemental que je vise en particulier, mais j'estime, de manière générale, que nos procédures sont trop lentes. Ce n'est en aucun cas une attaque contre le Sénat ou l'Assemblée nationale. Je fais simplement le constat

L'un des objectifs du projet de loi PACTE serait de faciliter la création d'entreprise. Selon vous, monsieur le ministre, l'un des obstacles à cette création résiderait dans les démarches à effectuer et la multiplicité des intervenants, due au nombre trop important de CFE répartis sur tout le territoire- près de 1 400 selon l'étude d'impact. Pour notre part, nous pensons que les obstacles à la création d'entreprise sont d'une autre nature, que votre projet de loi n'aborde pas. C'est d'un accompagnement véritablement pédagogique dont les aspirants entrepreneurs ont besoin : choix de la structure et du nom de l'entreprise, désignation des premiers dirigeants, détermination du siège social, réglementation de l'activité sous-jacente, options comptables et fiscales. Ces aspirants sont aussi en demande d'informations sur les entreprises récemment créées : quels sont les secteurs porteurs ? Quel est le pourcentage d'entreprises qui survivent au-delà de la première année ? Quels sont les retours d'expérience des entrepreneurs ?

ou d'une activité peuvent déjà être effectuées en ligne aujourd'hui. Les CFE restent des interlocuteurs clairement identifiés. Ces centres physiques permettent un accompagnement effectif des créateurs d'entreprise. Les supprimer en les substituant par une procédure entièrement dématérialisée est donc inacceptable, et ce d'autant que, à la suite de l'examen du texte à l'Assemblée nationale, seul un accompagnement facultatif à la vie de l'entreprise est proposé. À jour, nous ne savons toujours pas si le guichet unique sera à 100 % public. Encore une fois, sous couvert de simplification, une certaine privatisation des missions publiques se profile, ainsi qu'une déshumanisation des rapports administratifs. Ce que dessine ce projet de loi, c'est le démantèlement d'un service public, présent dans tout le territoire, de la création d'entreprise en France. Quel

engagés dans un débat politique respectueux : je ne me permettrais pas de vous traiter de rétrograde, d'ultralibéral ou de je ne sais quoi encore ! Pourquoi y aurait-il des modernes et des anciens ?

Mme Cathy Apourceau-Poly. L'article 1 du projet de loi vise à rendre obligatoires les formalités de création, de modification ou de cessation d'activité des entreprises par voie électronique. Au-delà de la remise en cause des réseaux d'accompagnement existants, cette obligation nie le fait que 8 millions de Français vivaient sans connexion internet en 2016, et que la fracture numérique est encore une réalité dans notre pays, notamment dans les

contre 31,2 % dans les zones rurales. Selon une étude de l'UFC-Que choisir, le déploiement de l'internet très haut débit laisse de côté une part croissante du territoire français 11,1 % des consommateurs sont désormais inéligibles à un internet de qualité, soit un débit supérieur à 3 mégabits par seconde. Ceux-ci vivent majoritairement dans de petites communes.

de loi. Cela pourrait éventuellement remettre en cause le monopole que vous essayez de créer en lieu et place des réseaux consulaires existants. Cela pourrait peut-être remettre en cause votre volonté d'asphyxier les chambres de commerce et d'industrie- les CCI -, de les étrangler, de les vider de leur substance, ce qui aboutira, en matière économique, au phénomène auquel nous assistons en matière d'organisation territoriale, à savoir une métropolisation de la réponse et, donc, un abandon de pans entiers du territoire national. Enfin, cette obligation ne risque-t-elle pas d'avoir comme effet,

l'amendement n° 97 rectifié. Pour notre part, nous sommes favorables au guichet numérique unique pour simplifier les démarches des entreprises lors de leur création, leur transformation ou leur cessation. la dématérialisation ne doit pas être une fin en soi. C'est pourquoi ce dispositif doit s'accompagner d'un certain nombre de garanties. Parmi celles-ci, la nature juridique du guichet unique et de l'organisme qui en aura la gestion est un enjeu central. À l'Assemblée nationale, monsieur le ministre, vous avez rejeté les amendements destinés à préciser ce point, qui est pourtant tout sauf anecdotique, et ainsi refusé de garantir dans la loi le caractère public de l'organisme qui sera mis en place. ailleurs indiqué qu'une mission d'information travaillait sur ce sujet. C'était en octobre 2018. Depuis, le flou persiste sur les intentions du Gouvernement. Vous avez notamment indiqué à l'Assemblée nationale que vous n'excluiez pas de faire appel à un opérateur privé. En tout état de cause, nous arrivons à un stade de la navette parlementaire où le Gouvernement doit clarifier ses intentions. Pour notre part, elles sont claires : nous proposons d'inscrire dans la loi que l'organisme sera de nature publique,

Pourtant, il ne nous paraît pas sain de confier à un opérateur privé une mission qui relève de la puissance publique, surtout lorsqu'il s'agit de garantir le maintien d'un service dont on vient de rappeler l'importance, de garantir l'égalité de traitement, la neutralité, l'adaptabilité et la mutabilité du dispositif, conformément à ce qui fonde la conception française du service public, et ce d'autant que la question de la protection des données est aussi fondamentale. Mais lorsque l'objectif visé reste de réaliser des économies- 23 millions d'euros par an grâce aux effets de mutualisation et d'échelle -, ces questions pourtant essentielles passent au second plan

Je crois savoir que la concision est une qualité, mais que la précision en est une autre. Très franchement, la chose irait mieux en l'écrivant.

Cet amendement reprend une position exposée lors de l'examen du texte en commission à l'Assemblée nationale. Il est en effet important de préciser que la création d'un organisme unique doit pouvoir être gérée par l'État d'une part, parce que les documents peuvent contenir des informations privées ; d'autre part, parce que l'externalisation de services implique quasi systématiquement une augmentation des coûts pour les finances publiques et une réduction de la qualité des services offerts aux usagers. Or l'État est parfaitement en capacité de gérer

Il prévoit que les dossiers déposés ne sont réputés réguliers et complets, et par conséquent juridiquement conformes, qu'à partir du moment où l'ensemble des organismes destinataires- les services fiscaux, les URSSAF, les caisses sociales, les répertoires des métiers et les registres du commerce et des sociétés -ont pu en contrôler la régularité ou en apprécier la validité, conformément à leurs missions. En effet, l'accusé de réception envoyé par le guichet électronique ne doit pas pouvoir être considéré par le déclarant comme une validation légale avant que tous les organismes aient été en mesure de contrôler le dossier. Il s'agit

: La parole est à M. Maurice Antiste. Cet amendement vise à sécuriser les déclarations des entreprises déposées auprès du guichet électronique unique, en garantissant aux futurs entrepreneurs la régularité de la validation de leur dossier. que l'accusé de réception émis par le guichet unique soit considéré comme une validation légale après que tous les organismes ont pu contrôler le dossier. Durant ce laps de temps, l'entrepreneur pourrait recevoir

? Prévoir que le dépôt ne vaudrait déclaration que lorsque le dossier est régulier et complet au regard des règles applicables aux formalités à accomplir auprès de tous les organismes destinataires concernés constituerait un retour en arrière par rapport à la simplification apportée depuis 1994 en matière de formalités administratives des entreprises. En outre, prévoir dans cet article la vérification du dossier par les destinataires des formalités est inutile : les dispositions en cause concernent uniquement la phase de dépôt des dossiers, et ne remettent pas en cause l'étape de contrôle de la validité des pièces fournies, qui bien sûr continuera à incomber aux organismes destinataires. L'avis est donc défavorable sur les deux amendements.

dans lequel vous pourrez déposer l'intégralité de vos déclarations. La première étape est la validation du dossier : une fois toutes les pièces déposées, le guichet unique vous informera que votre dossier est complet.

Ce document permettrait à ces entreprises de ne pas prendre de retard dans leurs démarches auprès de divers organismes, notamment les banques. Plus détaillé qu'un simple récépissé, ce document permettrait de porter à la connaissance des tiers un certain nombre d'informations figurant dans la demande d'immatriculation. Il ne s'agit pas là d'une amélioration accessoire car si, en effet, l'extrait Kbis définitif est généralement délivré au bout d'une semaine, ce délai peut parfois exploser. C'est notamment le cas outre-mer, en particulier à La Réunion, où la délivrance de ce document peut prendre jusqu'à six mois.

dont il n'est pas assuré qu'il permette à lui seul d'effectuer des démarches, dans la mesure justement où seule l'immatriculation définitive, par exemple au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, fait naître des conséquences juridiques effectives. Je demande donc le retrait de

et de rendre obligatoire la déclaration par voie électronique de la création d'une entreprise, au détriment des personnes qui éprouvent des difficultés avec les outils numériques. Il est proposé en conséquence que le décret précise les modalités de dérogation au dépôt par voie électronique pour les publics concernés.

le redis, le dispositif entrera en vigueur de façon progressive jusqu'en 2023, ce qui donnera le temps de détecter les difficultés d'accès au guichet de certains acteurs économiques. Il semble prématuré de prévoir d'ores et déjà des dérogations.

le site internet, elle se rendra dans la CCI, où nous avons prévu que serait maintenue la possibilité du dépôt physique de la candidature. Ensuite, l'agent de la CCI

on demande d'utiliser un outil dont les conditions d'utilisation ne sont pas aujourd'hui assurées.

En même temps, on nous dit : même si vous n'êtes pas desservis pour l'instant, vous devrez tout de même utiliser les moyens électroniques existants,

par voie électronique les dépôts, notamment de dossiers de création d'entreprise. La vérification qui sera opérée à ce stade se limitera à la complétude du dossier et à la régularité des pièces produites, mais il ne reviendra pas à cet organisme unique de contrôler la qualification professionnelle éventuellement

telles que les déclarations d'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise, l'ACCRE, les enregistrements des contrats d'apprentissage, l'enregistrement des fonds agricoles. Certaines chambres d'agriculture proposent des prestations complémentaires souvent indispensables au service public, permettant aux agriculteurs de bénéficier d'un accueil personnalisé et adapté à leurs difficultés : diagnostic du dossier, aide aux réponses au formulaire par téléphone ou en rendez-vous, information sur les renseignements à fournir, contrôle de conformité de l'imprimé rempli ... La liste est loin d'être exhaustive. Elles vérifient aussi la cohérence entre la déclaration et la situation connue de l'entreprise, les pièces justificatives et les renseignements fournis. Ainsi, elles assurent ce qui fait défaut à votre dispositif, un accompagnement personnalisé adapté aux difficultés rencontrées par les agricultrices et les agriculteurs. C'est l'essence même du service public de proximité

En effet, la suppression programmée des CFE, et notamment ceux des chambres d'agriculture, entraîne la suppression du recours aux informations qu'ils détiennent dans le cadre de vérifications administratives liées au contrôle des structures des exploitations agricoles. la fin des CFE, nous perdons une source pertinente de vérification des informations déclarées par les demandeurs d'autorisation d'exploiter. Cet amendement vise donc à

prévoit d'étendre les vérifications administratives en permettant également la consultation du registre des bénéficiaires effectifs. Cela permettrait, dans un second temps, de se prémunir contre certains montages avec pluri-participations dans les sociétés qui viseraient à contourner la législation des structures agricoles. Cet amendement a donc un double objectif : assurer une meilleure cohérence des textes et garantir davantage de transparence dans les transactions sociétaires agricoles. Quel

n° 562, la création du guichet électronique unique et la disparition progressive des CFE des différents réseaux constitueront une simplification pour l'ensemble des entrepreneurs, y compris dans le domaine agricole. Les réseaux consulaires resteront intégrés dans la procédure de dépôt et continueront d'assurer les mêmes fonctions qu'aujourd'hui

! Tous ceux qui croient ici à l'entrepreneuriat, à la simplification et à l'accélération des procédures, mais aussi au conseil physique pour ceux qui en ont besoin devraient donc se réjouir de ces propositions et accepter le texte tel qu'il est. L'avis est donc défavorable

La fracture numérique en outre-mer est beaucoup plus profonde que dans l'Hexagone, notamment dans les départements de la Guyane et de Mayotte. L'article 1 de ce projet de loi risque de l'alourdir encore en limitant les possibilités de création d'entreprise pour les personnes situées dans les zones non ou mal couvertes par l'internet haut débit. L'effet de la réforme serait alors contre-productif en éliminant de la compétition économique ceux qui résident dans les régions isolées, comme les communes de l'intérieur de la Guyane, et mal équipées, alors que ce sont justement celles qui ont le plus besoin de développement. Cet amendement vise donc à attendre la fin, prévue en 2022, du plan France très haut débit, dont dont l'objectif est la couverture intégrale du territoire en connexion internet à très haut débit, avant de rendre obligatoire en outre-mer la procédure dématérialisée de création d'entreprise.

mais il est douteux que le Gouvernement mette en place le guichet unique électronique avant cette date si les conditions techniques d'accès du plus grand nombre des acteurs économiques ne sont pas garanties. La modification proposée à travers l'amendement semblant inutile, l'avis est défavorable.

compte tenu de la situation financière des CCI, de supprimer dès 2021 les CFE qu'elles gèrent. Le report sur les CFE des autres réseaux devrait être d'autant plus limité que le guichet unique électronique absorbera la majeure partie des démarches des entrepreneurs effectuées auprès des CFE des CCI.

Les présidents et les organisations des chambres de commerce sont en train de mettre en oeuvre ces plans. Si l'on garde ces personnels, alors même qu'ils partiront dans quelques mois et qu'ils ont des opportunités, il faudra les remplacer

De fait, la mise en place d'un guichet numérique qui peut apparaître comme une mesure de simplification au niveau national risque de créer une nouvelle inégalité en outre-mer. Nous avons entendu votre position sur Cet amendement vise donc à demander que soient évalués spécifiquement les effets de la mise en oeuvre d'une telle mesure au sein des territoires d'outre-mer. prévoit que, dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à l'impact en outre-mer de la mise en oeuvre du dispositif de guichet unique au sein des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

concernant ces dernières. Il s'agit de mettre en place une centralisation des informations destinées à identifier les personnes physiques ou morales qui exercent une activité économique et à diffuser les informations recensées. Il faut noter qu'en plus de la nécessaire transparence en matière commerciale, ces répertoires permettent la réalisation de statistiques et de recherches. Selon l'étude d'impact, dans le cas du fichier SIRENE par exemple, il est précisé que celui-ci « constitue une référence servant de base pour toutes les investigations statistiques sur les entreprises, enquêtes ou exploitations de sources administratives. Il est utilisé notamment pour tirer les échantillons des enquêtes annuelles d'entreprises dans l'industrie, la construction, le commerce et les services. Le Gouvernement serait également habilité dans le même délai à simplifier par voie d'ordonnance les obligations déclaratives des entreprises et les modalités de contrôle des informations déclarées, ce qui n'est pas rien à l'heure où l'opacité semble de mise. Or le flou est total puisqu'il semble que les informations centralisées seraient ensuite dispatchées aux différents organismes qui continueraient à avoir leur propre fichier. Il ne s'agirait en fait que de la création d'un énième fichier puisque, selon l'article 2, ce registre général se substituera « à tout ou partie » des registres existants. De plus, selon l'étude d'impact, la réforme pourrait avoir des incidences organisationnelles, techniques, financières et humaines pour les teneurs des registres actuels. Mais il n'est pas possible à ce stade de décrire ces incidences. La représentation nationale devra attendre et voter un blanc-seing. Pourtant, comme vous l'avez rappelé, monsieur le ministre, ce registre unique, ce sera « des millions de données et de situations à traiter ». Or nous ne savons pas à qui il sera confié. Que

Pour toutes ces raisons, nous souhaitons que ce sujet fasse l'objet d'un texte dédié et non pas d'une habilitation, de surcroît de deux ans. votre amendement fait référence à la substitution de tout ou partie des répertoires et registres, c'est-à-dire à la version de l'article 2 tel qu'adopté par nos collègues députés.

teneurs de registre, il n'y a pas à proprement parler d'instruction de l'administration. Le terme de « délai de traitement », que la commission spéciale a adopté, est plus large et englobe tous les cas de figure. Ainsi, quelles que soient la forme et la nature juridique du futur registre, la formule pourra s'appliquer.

Je comprends parfaitement l'argumentaire de Mme la rapporteur, mais étant par nature favorable à la réduction des délais administratifs et à l'accélération des procédures au service des entrepreneurs, je m'en remets à la sagesse du Sénat.

importants. D'abord, nous avons précisé les registres concernés par la fusion, alors que tel n'était pas le cas dans le texte qui vous avait été transmis. Il s'agit de tous les registres et répertoires d'entreprise existants, locaux et nationaux, à l'exception des registres du commerce et des sociétés locaux et des autres registres qui sont tenus par les greffiers des tribunaux de commerce, ainsi que du répertoire SIRENE, tenu par l'INSEE. Je le redis, grâce au travail que nous avons fait ensemble, madame la rapporteur, le champ est précisé et les registres concernés figurent

En effet, ils sont les garants de la conformité des informations qui seront désormais centralisées, et notamment la légalité de l'installation, le contrôle de l'absence d'interdictions et le contrôle de la qualification professionnelle. La parole est à M. Yvon

L'article 2 tend à la création d'un registre général des entreprises ayant pour objet la centralisation et la diffusion des informations les concernant. Il prévoit le maintien du contrôle de ces informations avant leur centralisation et leur diffusion par les officiers publics et ministériels. Dans le même objectif, il est indispensable également que le rôle des teneurs des registres publics existants, pour les activités relevant de leurs compétences, soit maintenu. En effet, les registres publics existants sont les garants de la conformité de ces informations, notamment la légalité de l'installation, le contrôle de l'absence d'interdictions et le contrôle de la qualification professionnelle. Quel est l'avis de la commission

Désormais, les intentions sont à la fois plus claires et plus « sécurisantes ». Elles sont d'abord plus claires, car seuls le répertoire SIRENE tenu par l'INSEE et les registres locaux tenus par les greffiers des tribunaux de commerce ou équivalents seront maintenus. Le premier est conservé pour des raisons de connaissances statistiques et les seconds afin d'éviter un risque juridique et financier pour l'État, comme cela est indiqué dans l'étude d'impact.

pour le suivi des professions et le contrôle des qualifications avaient fait part de leur inquiétude pour ce qui concerne l'accès aux informations du nouveau registre. Or il est ici prévu que les chambres consulaires disposent d'un accès gratuit et permanent aux informations contenues dans ce registre. Elles pourront donc continuer à opérer les contrôles nécessaires et les missions d'accompagnement sans difficulté, et obtenir les informations utiles pour les professions concernées. Compte tenu de ces améliorations, je propose de donner un avis favorable

question des quotidiens, voire des hebdomadaires, qui sont habilités à publier des parutions légales et judiciaires.

l'aggravation de ce phénomène ne tient pas tant à une diffusion plus importante des informations qu'à une défiance généralisée à l'égard de nos médias. Le réflexe logique aurait donc été de réinvestir massivement dans la presse pour lui redonner du cachet, d'un investissement d'État global pour garantir le pluralisme de la presse. L'aide au développement de ressources propres des titres est le seul moyen permettant à terme de lutter efficacement contre la concentration de toute la presse dans quelques mains. Le bilan est aujourd'hui clair l'État se désengage massivement des aides à la presse privée et retire ses subsides à l'audiovisuel public. On aurait donc pu se dire que l'objectif était de pousser les titres à développer des ressources propres. Mais cela était sans compter avec la volonté du Gouvernement toujours plus loin en matière de réduction des coûts des entreprises. Le résultat est illustré par cet article 3, qui revient sur un des principes fondateurs des annonces judiciaires et légales : la tarification à la ligne. Cela tient pourtant du bon du bon sens : plus une entreprise prend de place dans le journal, plus elle paie. Cela compense à la fois l'espace occupé que la publication ne pourra pas utiliser et les retombées économiques attendues par l'entreprise en question. Ce système, c'est ce qui permet à des dizaines de titres de presse, notamment locaux et spécialisés, de survivre. Cela permet d'ailleurs à des entreprises extra-spécialisées d'avoir accès à une audience que l'on sait intéressée sur le principe aux activités de l'entreprise. On est donc dans un modèle gagnant-gagnant. Mais la tarification forfaitaire voulue par le Gouvernement vient mettre à bas ce principe, avec des coûts déjà estimés à 18,5 millions d'euros pour ces titres. Il s'agit d'un nouveau coup porté aux éditeurs de presse, après la baisse des aides et l'instauration de la taxation spécifique destinée à sauver Presstalis. Certes, le Gouvernement a acté un lissage de la mesure sur cinq ans pour permettre d'amortir quelque peu les pertes pour les titres. Il n'empêche que l'on parle à plus ou moins long terme de plusieurs millions d'euros de pertes que le Gouvernement n'entend pas compenser. Et quand bien même l'aurait-il fait, l'on est en droit de s'interroger : pourquoi les entreprises ne devraient-elles pas payer à leur juste valeur un service sur lequel elles font des bénéfices réels, notamment en termes de visibilité ? Quel

n'ont pas remis en cause cette évolution. L'avis est donc défavorable.

avec la presse, en particulier avec la presse quotidienne régionale et la presse hebdomadaire régionale. Nous avons trouvé un équilibre : après avoir envisagé la possibilité d'une suppression totale des annonces légales- c'était, dans un souci de simplification,

habilitée à publier des annonces judiciaires et légales, édite la plateforme centrale numérique actulegales.fr, agréée par les ministères de la justice et de la culture. Cette plateforme numérique diffuse, à destination du grand public et des acteurs économiques territoriaux, une information économique de première importance, constituée de l'intégralité des annonces judiciaires et légales relatives à la vie des sociétés, publiées quelques jours

et fait peser une charge supplémentaire de 91 millions d'euros par an sur les entreprises, alors que les journaux d'annonces légales remplissent déjà la mission de publication avec un délai de publication plus court de vingt-trois jours. Maintenir ce doublon nuit aux objectifs du projet de loi PACTE : simplifier et réduire le coût de la création d'entreprise. Monsieur le ministre, lors des débats en première lecture à l'Assemblée nationale, vous avez indiqué qu'il fallait faire en sorte de n'avoir plus qu'une seule comptabilité des opérations économiques dans le pays, au lieu de deux.

actualisée à plusieurs reprises, qui leur assigne la mission de publier les annonces judiciaires et légales, les AJL. Qu'elle soit d'information politique et générale, économique, agricole ou judiciaire, cette presse de proximité est lue par près de trente millions de lecteurs français, qui ne disposent pas encore d'un accès numérique suffisant. les JAL, irriguent donc l'ensemble des circuits économiques des territoires français, en participant à la transparence du monde économique. Le modèle économique de ce secteur a été gravement bousculé par l'évolution technologique et les modes de consommation de l'information- gratuité, mobilité, etc -, auxquels la crise économique a ajouté son lot de difficultés- régression de la publicité, alourdissement des charges sociales, investissements de survie. L'ouverture de la publication des AJL aux services de presse en ligne ainsi que l'extension de la tarification au forfait de ces annonces auront un impact inégal sur les journaux habilités à publier des annonces légales. En effet, les JAL sont composés majoritairement d'entités économiques de petite taille aux moyens limités et morcelées sur l'intégralité du territoire national. La nécessaire mutation de leur modèle économique requiert un délai suffisant d'adaptation afin de mieux préparer cette transition et d'éviter la disparition des plus fragiles, ainsi que des emplois concernés.

d'avoir un complément d'information qu'ils n'auraient pas forcément dans le journal habituel, unique. J'ajoute que ces annonces judiciaires de proximité

à lui. Il ne faut pas que nous lui enlevions cela, d'autant que notre demande est tout de même facile à satisfaire : il s'agit juste de laisser un peu de temps à ces journaux pour s'adapter. C'est le même paradoxe que précédemment : on demande,

le nombre de lecteurs ou d'utilisateurs des connexions internet potentielles qui n'existent pas suffisamment et qui ne couvrent pas tout le territoire ? Il y a là une espèce de contradiction, et la solution facile,

? La commission spéciale s'est déjà prononcée sur cet amendement. Je le rappelle, l'impact de la mesure sera très progressif, puisque le Gouvernement a annoncé que l'évolution tarifaire serait étalée sur cinq ans, ce qui laissera le temps aux journaux de s'adapter économiquement. Par ailleurs, l'ouverture à la presse en ligne ne va certainement pas bouleverser leur modèle économique du jour au lendemain. Le Syndicat de la presse indépendante d'information en ligne a d'ailleurs indiqué que seul un tiers des éditeurs qu'il représente, c'est-à-dire une cinquantaine, a des titres ayant vocation à publier des annonces judiciaires et légales.

le stage préalable à l'installation des artisans, que le Gouvernement souhaitait initialement supprimer, est un outil indispensable à la réussite des projets des entrepreneurs, à la diffusion des bonnes pratiques et à la pérennité de l'activité. comporte, dans un premier volet, une initiation à la comptabilité générale et à la comptabilité analytique, ainsi qu'une information sur l'environnement économique, juridique et social de l'entreprise artisanale. Ce stage porte aussi sur la responsabilité sociale et environnementale, ce qui est à mon sens essentiel pour l'entreprise de demain- celle que vous avez appelée « l'entreprise du XXI siècle qu'elle soit artisanale, agricole ou commerciale. Un second volet comprend une période d'accompagnement, postérieure à l'immatriculation du créateur ou du repreneur d'entreprise au répertoire des métiers ou au registre des entreprises formation et accompagnement, c'est aussi de cela que les entrepreneurs ont besoin. C'est pourquoi nous ne comprenons pas que, sous couvert de simplification et d'économie, ce dispositif, qui a été modifié seulement en 2016, soit déjà remis en cause, d'autant que, à trois ans, les entreprises dont les créateurs

Si la commission a réintroduit une obligation de stage allégée, il n'en demeure pas moins qu'elle maintient la suppression d'un encadrement, par la loi, du prix de ce stage. Cela aura évidemment évidemment pour effet de libéraliser les offres de formation, dont les prix pourront devenir exorbitants, ... Pourquoi ? ... alors même que l'une des raisons évoquées pour supprimer ou modifier le dispositif était son coût trop élevé

La nouvelle rédaction de celui-ci, issue des travaux de la commission, sur l'initiative de notre rapporteur, me semble parfaitement équilibrée. En effet, cette formation permet de rappeler au créateur d'entreprise les notions fondamentales et minimales qui lui seront indispensables pour gérer son activité. présente donc une réelle utilité, surtout pour les anciens ouvriers qui disposent de compétences techniques solides, comme cela a été rappelé à l'instant, mais qui n'ont pas forcément les connaissances requises en matière de gestion d'entreprise. Avec cet article, l'objectif du Gouvernement, qui va défendre dans un instant son amendement n° 256, est de rendre plus simple la création d'entreprise, et de laisser le choix à chaque créateur d'opter pour un accompagnement adapté. On peut comprendre cet amendement, mais il faut quand même savoir et avoir à l'esprit que, selon l'étude d'impact, le gain moyen sera de 242 euros pour un micro-entrepreneur et de 548 euros pour un artisan choisissant un autre statut. Ces chiffres sont toutefois à mettre en parallèle, ce qui me paraît infiniment plus important,

compte tenu des taux que je viens de citer, constituerait un facteur de concurrence déloyale ; en maîtrisant mal leur rentabilité, les créateurs ont tendance à pratiquer des prix trop bas, néfastes pour leur secteur. On crée donc là,

l'activité des chambres de métiers en termes de stages, mais la réussite des femmes et des hommes qui osent se lancer dans la vie économique et monter leur entreprise. Nous sommes un certain nombre à avoir pris le temps-

mais il y a tous les autres, qui en ont absolument besoin. Parfois- c'est arrivé -, il faudra dissuader certaines volontés de créer leur entreprise parce qu'elles ne sont pas prêtes.

certes, mais les chambres de métiers y tiennent beaucoup et ils sont absolument utiles. L'accompagnement de la création entreprise est quelque chose d'essentiel.

tous ceux qui ont déjà suivi un accompagnement à la création d'entreprise ou tous ceux qui ont une formation au moins égale au niveau du stage ; il ne reste donc vraiment

et social de l'entreprise et sur la responsabilité sociale et environnementale de celle-ci. Est-il sérieux de balayer en une journée tous ces sujets, pour quelqu'un

ils étaient unanimes sur le fait qu'il fallait absolument maintenir ce stage. Bien entendu, ils n'y étaient pas forcément favorables au préalable

modifier les choses, les améliorer, notamment sur la question du droit bancaire, sur la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise, sur un certain nombre de droits. On peut renforcer ce stage, mais on ne peut pas le rendre facultatif, il faut que ce soit obligatoire. Mon deuxième point

des opérateurs publics

Le président Pompidou avait proposé un stage facultatif, qui a été rendu obligatoire par François Mitterrand. Tout cela est parfaitement démocratique. Je suis simplement surpris de voir désormais Les Républicains du côté de François Mitterrand et des socialistes.

de la confiance que je fais aux jeunes artisans qui ont leur qualification et qui sont prêts à se lancer dans la vie, au nom du sens des responsabilités, qui nous conduit à maintenir la possibilité, pour tous ceux qui le souhaitent,

le but. J'admire également la hauteur des arguments que vous avez avancés : je n'ai toujours pas bien compris les raisons pour lesquelles vous vous opposez à la formation des artisans.

argumenté contre une « économie administrée ». Je suppose que vous ne savez pas ce que c'est ! Vous employez des mots dont vous ignorez la signification. Je suis socialiste, et je peux vous dire que nous avons parfaitement respecté l'économie de marché au cours des différentes alternances. Vous n'avez d'ailleurs sans

le ministre, ceux qui seraient « archaïques » et ceux qui seraient « nouveaux ». Le « nouveau monde » rejette dans les limbes tous ceux qui auraient la tentation de dire qu'on peut conserver un certain nombre de choses et que le changement ne porte pas en lui une vertu.

Ce stage, qui peut sembler inutile à vos yeux, permettra à des personnes qui veulent s'installer de s'insérer dans un corps professionnel, ou du moins dans une identité professionnelle. La proposition de la commission, qui considère qu'il faut conserver un stage, quitte à le faire évoluer, permet de continuer à considérer qu'on administre bien que de près et que les corps intermédiaires ont véritablement un sens dans notre économie.

nous avons tous besoin de plus de formation. Il faudrait d'ailleurs, monsieur le ministre de l'économie et des finances, que la majorité des Français soient mieux sensibilisés aux questions économiques, ce qui permettrait peut-être

à s'inscrire dans des parcours de formation et à faire en sorte d'être encore plus performants, en ajoutant à la connaissance technique du métier une compétence technique de chef d'entreprise.

et que je reste convaincu qu'on peut devenir artisan sur la base de la qualification qu'on a obtenue, sans être obligé de passer par ce stage. Je ne partage donc pas les arguments qui ont été développés ici, tout en concevant parfaitement qu'on puisse demander,

en revanche, que je ne les ai pas présentées, monsieur le sénateur. Première raison : j'estime que ce dispositif est injuste- 40 % des artisans qui s'installent, au nom de la liste que je vous recommande de lire, échappent à ce stage obligatoire.

beaucoup de jeunes artisans qui voudraient s'installer, et qui ne pourront pas le faire dans des conditions adéquates. Pour reprendre la remarque de Michel Raison sur Pompidou, il faut arrêter d'emmerder les Français. En proposant la suppression du stage préalable à l'installation obligatoire, ce sont les jeunes artisans français qui veulent s'installer que je souhaite arrêter d'emmerder.

La séance est suspendue.